sécurité globale », dont l'examen a débuté hier à l'Assemblée. Il y pointe des atteintes importantes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'association et de réunion pacifique. Nous voilà en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l'homme. Vous en conviendrez, ce n'est pas un honneur Le rapport insiste notamment sur l'article 24, qui vise à interdire la diffusion d'images d'agents des forces de l'ordre non floutées, assortie d'une sanction de 45 000 euros d'amende et d'une peine d'un an de prison. Combien de violences policières échapperont-elles au radar de la justice ? Que deviendra la liberté de la presse et d'informer ? Monsieur le ministre, comment pouvez-vous laisser la France se renier comme patrie des droits de l'homme en appuyant cet

les termes de la loi que vous évoquez et ce fameux article 24 qui fait tant couler d'encre. J'observe que, dans les médias, les uns et les autres donnent leur point de vue sur cet article 24 sans toujours savoir exactement

: « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique,

La crise que traversent nos commerces, le financement du chômage partiel, les aides à nos petites et moyennes entreprises (PME) et aux ménages modestes, le renforcement de notre système de santé, la transition énergétique et numérique sont des enjeux majeurs et urgents. Or notre plan de relance dépend intrinsèquement de celui de l'Union européenne. La Hongrie et la Pologne ont posé leur veto au financement de l'avenir de l'Europe. Ils s'opposent à ce que 450 millions d'Européens, y compris leurs propres citoyens, bénéficient d'une relance rapide dont ils ont cruellement besoin. La raison en est le refus de s'engager à respecter l'État de droit. En Europe et au XXI siècle, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, le respect des droits fondamentaux servent de monnaie d'échange à des apprentis dictateurs adeptes de la démocratie illibérale. Ils préfèrent nous entraîner tous dans leur chute plutôt que de perdre la face dans leur pays. Monsieur le secrétaire d'État, la réussite rapide de ce budget européen est une nécessité. Le temps presse et la marge de manoeuvre paraît bien étroite.

a été adopté par le Parlement européen, après quelques semaines de négociations avec les différentes institutions européennes. Je tiens à préciser que, par rapport à l'accord trouvé au mois de juillet, ce plan a été amélioré. Un certain nombre de priorités politiques essentielles pour la France, Erasmus, les programmes de financement de la recherche- y compris des vaccins -, ou le financement de notre coopération en matière sanitaire, avaient vu leurs crédits augmenter, pour un total de 16 milliards d'euros. À la suite de cet accord entre institutions, deux pays ayant pourtant suivi jour après jour les négociations ont fait état de leur volonté de bloquer l'ensemble de

Précision encore plus importante, cela ne remettra pas en cause- je le dis sous le contrôle du ministre chargé de la relance -le plan de relance de 100 milliards d'euros. Bien que plus de 40 milliards d'euros soient apportés par l'Union européenne, cela ne ralentira pas

M. Pierre Médevielle, pour la réplique. Monsieur le secrétaire d'État, nous ne pouvons que vous souhaiter un plein succès dans les négociations à venir, d'autant qu'il semblerait que la Slovénie ait rejoint la Hongrie et la Pologne.

mais les commerçants de proximité attendaient de votre part une annonce pour une reprise le 12 novembre dernier. Vous leur avez donné rendez-vous dans quinze jours, pour le 1décembre. Ce lundi, Bruno Le Maire prédit des réouvertures dès le 27 novembre le lendemain, le ministre de la santé ne voit pas les conditions réunies pour une réouverture des commerçants le 27 ; ce même mardi, c'est-à-dire hier, Gabriel Attal indique que le Gouvernement tranchera « la semaine prochaine

On ne peut ajouter à la crise sanitaire, économique et sociale une crise humaine qui pointe avec le désespoir de certains. Monsieur le Premier ministre, vous devez en tenir compte ! Pourquoi laisser fermés les commerces de proximité ? Est-ce vraiment pour éviter un trop grand flux de clients entre les différents commerces ? Aucun élu, dans cet hémicycle, ni vous-même, ne peut imaginer que, dans les coeurs de ville, les centres-bourgs et les quartiers, l'affluence de clients masqués serait telle chez les commerçants qu'elle impliquerait On mesure l'iniquité de traitement avec d'autres formes de commerce et avec, notamment, les transports en commun, où la promiscuité est sans commune mesure. En réalité, aucune raison scientifique ni donnée statistique ne nous a jamais été fournie pour justifier ces fermetures. La prévention peut être revue, les protocoles renforcés alors que beaucoup a déjà été fait en dialogue avec les commerçants et, en particulier, les restaurateurs qui ne demandent qu'à travailler ! Monsieur le Premier ministre, ma question est simple : à quelle date pourront-ils rouvrir ?

votre connaissance du terrain, votre proximité avec les petits commerces- notamment ceux de Tours, mais sans doute aussi ceux de toute la France -, pour savoir que vous comprenez parfaitement ce que vous dites ne pas comprendre. Vous comprenez parfaitement que notre préoccupation à tous, ici, celle du Premier ministre, celle du Gouvernement et, je pense, celle de toutes les sénatrices et de tous les sénateurs, c'est de garantir la sécurité sanitaire des Français

dans l'intérêt des commerces et dans l'intérêt des Français dans leur ensemble.

À quelques semaines de l'ouverture de la saison d'hiver, les acteurs et territoires touristiques sont extrêmement inquiets. Ces acteurs et territoires sont variés : on pense tout de suite au secteur de la montagne, mais n'oublions pas l'outre-mer, qui accueille, en cette saison et en temps normal, de nombreux métropolitains. La montagne La montagne et les territoires ultramarins ont, bien sûr, des problématiques touristiques distinctes. Côté outre-mer, des territoires comme la Polynésie française ne bénéficient pas du dispositif de chômage partiel applicable en métropole. monsieur le secrétaire d'État, comment comptez-vous préserver l'emploi et soutenir spécifiquement les entreprises de tourisme ultramarines ? Côté montagne, la fermeture, le 15 mars dernier, des 350 stations, avait amputé la précédente saison d'hiver de 20 %. Les enjeux de la prochaine saison sont d'une tout autre ampleur puisque c'est l'intégralité de la saison qui est menacée, ce qui représente 10 milliards d'euros de retombées économiques, 10 millions de vacanciers, 120 000 emplois directs, 360 000 emplois indirects et leurs familles, ainsi que notre place de troisième destination mondiale de ski. Restreindre l'accès aux stations serait une catastrophe. Les professionnels de la montagne ont pris leurs responsabilités, et vous le savez. Ils élaborent, avec les services de l'État et les maires, un protocole sanitaire spécifique, qui doit être validé dans les meilleurs délais pour limiter les dégâts. Monsieur le secrétaire d'État, avez-vous une idée du calendrier de sa mise en oeuvre ? Par ailleurs, pour sauver la saison d'hiver, les classes de neige vont être déterminantes, en particulier pour les stations-villages. Êtes-vous en liaison avec le ministre de l'éducation nationale pour faire en sorte que les séjours scolaires ne soient pas annulés et que des instructions claires soient données en ce sens au rectorat ?

projet élaboré par le cabinet Accenture -, la possibilité d'une reprise par un fabricant de pneumatiques extraeuropéen focalise les espoirs des 863 salariés du site de Béthune et de leurs familles.

que quatre manifestations d'intérêt ont déjà été enregistrées. Vos services nous ont confirmé que, pour l'une d'entre elles, nous en étions déjà au stade de la prise de rendez-vous. La perspective de l'établissement de quotas d'importation à l'échelle européenne est un facteur, semble-t-il, favorable à l'activité de nouveaux producteurs. Je ne fais pas confiance à Bridgestone pour mener, à terme, un projet de reprise fiable, d'autant que le temps est compté. C'est pour cette raison que je vous demande, madame la ministre, un engagement : Bridgestone doit céder le site pour un euro symbolique. Le directeur béthunois de l'entreprise a déclaré être prêt à examiner la demande de remboursement des aides publiques perçues. Je vous demande de l'y contraindre. À ce stade préliminaire de la recherche d'un repreneur, je n'attends pas de vous la liste nominative des entreprises intéressées. Mais pouvez-vous nous préciser les critères qui vous amèneront à valider un projet par un producteur de pneumatiques ? La parole est à Mme la ministre

pourtant rentable, mais peut-être pas suffisamment, que nous avions construit avec Accenture et les élus du territoire. Je veux vous le dire : le combat n'est pas terminé. Comme vous l'avez indiqué, nous continuons à avoir des contacts étroits

Enfin, nous allons continuer à travailler et à nous battre pour que les conditions de revitalisation de ce territoire soient à la mesure des moyens de Bridgestone. Vous avez raison de dire que nous devons être exigeants avec la direction de Bridgestone. J'ai été très claire avec ses

Ce passage contraint et massif au télétravail ne doit toutefois pas servir de référence à une diffusion plus large de ce mode de travail. Le télétravail en situation de crise n'est pas représentatif d'un télétravail efficace et équilibré. et équilibré. Comme tous les modes d'organisation, il doit être pensé et structuré, requérant en outre une formation préalable, des outils adaptés, un partage de l'information à l'abri des menaces cyber, une réduction de la fracture numérique entre les territoires et de nouveaux processus dématérialisés. Le télétravail présente, à première vue, de nombreux avantages : sur le plan environnemental, en limitant les transports ; sur le plan territorial, en désengorgeant les métropoles et en libérant des surfaces ; sur le plan personnel, en apportant flexibilité dans la vie de nos concitoyens. Apparaissant, de prime abord, comme une petite révolution, il est avant tout une adaptation à une société qui évolue sans pour autant annihiler les bénéfices indiscutables d'un lien social, qui reste plus que jamais essentiel. Pour cela, il faudra veiller à une forme de justice dans son application, tous les métiers n'y étant pas éligibles et tous nos concitoyens n'étant pas égaux devant les compétences spécifiques qu'il requiert. Nous devons travailler, dès aujourd'hui, à l'articulation optimale entre télétravail et présentiel, en considérant le premier de manière qualitative plutôt que quantitative. dès à présent travailler sur les effets collatéraux du télétravail : droit à la déconnexion, à la prévention des conduites addictives et des traumatismes psychologiques. Au vu des nombreux enjeux de cette nouvelle pratique, n'est-il pas opportun, madame la ministre, de prévoir une grande réflexion autour de ce sujet majeur ? ? Quelle stratégie le Gouvernement souhaite-t-il mettre en oeuvre concrètement, afin de permettre à nos dirigeants comme à nos salariés d'appréhender ce virage sociétal avec succès ?

De fait, une partie importante de notre activité économique s'était arrêtée. Cette fois, nous avons voulu maintenir l'activité économique tout en posant des règles exigeantes en matière de télétravail. Cela fait maintenant deux semaines que ces règles s'appliquent. L'enquête que nous avons menée début novembre nous montre que, dans leur très grande majorité, les employeurs et les salariés jouent le jeu ; je les en remercie.

est sur un poste qui n'est pas du tout télétravaillable. Deuxième enseignement : l'enquête nous montre en outre que la très grande majorité de ceux qui peuvent télétravailler l'ont fait, et ils l'ont fait davantage que la semaine précédente. Troisième enseignement : le télétravail cinq jours sur cinq représente un véritable effort pour les salariés, qui peuvent parfois souffrir d'isolement. C'est le cas pour quatre salariés sur dix.

Au-delà, nous devons tirer tous les enseignements de cette expérience, pour que le télétravail joue pleinement son rôle, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, dans la lutte contre le virus. Enfin, il s'agit d'inscrire le télétravail comme une pratique durable, dans de bonnes conditions, pour les employeurs et pour les salariés. C'est précisément le sens de la concertation engagée entre les partenaires sociaux en vue d'un accord national interprofessionnel. Nous souhaitons tous, me semble-t-il, que cette concertation puisse aboutir rapidement. La parole

Monsieur le Premier ministre, 1 328 537 décès dans le monde, 46 273 en France : tel est le bilan à ce jour de la pandémie causée par la covid. Je n'oublie pas non plus les femmes et les hommes sortis de nos hôpitaux qui vivent aujourd'hui avec des séquelles. Permettez-moi, à cet égard, de remercier les personnels de santé de leur engagement sans faille, malgré le contexte plus que difficile. La crise planétaire affecte l'humanité tout entière sur les plans social, économique et démocratique. Pour autant, dans ce marasme, une lueur d'espoir vient de naître avec l'annonce, par plusieurs laboratoires, à disposition prochaine de vaccins efficaces. Il nous faut saisir cet espoir et nous y préparer. D'ailleurs, la priorité absolue définie dès le 9 juillet dernier par le conseil scientifique est d'anticiper et de disposer d'un plan national de vaccination.

sera disponible pour les Français ? Quels sont les publics prioritaires ? Quel sera le coût ? de la logistique et du calendrier de vaccination des Français ? Quelle est la mobilisation de la recherche française dans ce dispositif ? Quelle aide apporter aux pays en développement ? Enfin,

de l'ensemble des pays du monde, à l'arrivée d'un vaccin qui permettra de vacciner la population. Sur ce point, nous avons déjà avancé. Nous avançons avec prudence, parce que nous en sommes encore aux essais de phase III, avec des résultats

nos concitoyens. Il s'agit d'identifier des centres, des transporteurs, des conditions de transport, sachant que les différents vaccins ne nécessitent pas les mêmes conditions de stockage et de transport. À cet égard, nous travaillons sur plusieurs scénarios. Enfin, vous avez posé la question importante des publics cibles et prioritaires. Sur ce point, nous avons saisi la Haute Autorité de santé et le Comité consultatif national d'éthique, qui nous rendront leurs conclusions dans les prochains jours. C'est à la lumière de leur travail que nous serons en mesure de communiquer des informations sur ce sujet.

chargée de l'autonomie, l'état d'urgence sanitaire autorise les préfets d'outre-mer à placer en quarantaine ou à l'isolement toute personne arrivant sur leur territoire depuis une zone de circulation du virus. Depuis le début, j'ai défendu ardemment une sécurité sanitaire renforcée à l'entrée sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le 7 novembre dernier, après de nombreuses sollicitations, le préfet a décidé le placement systématique en quarantaine, suivi d'un second test PCR, de toute personne arrivant sur l'archipel. Ce dispositif permet d'identifier très tôt les cas suspects, de les isoler et d'éviter la circulation du virus. Le décret du 31 janvier 2020 prévoyait, dans sa première version, qu'une personne placée en quarantaine ou en isolement et pour qui le télétravail était impossible était prise en charge financièrement par l'assurance maladie au titre d'un arrêt de travail dérogatoire. Lors de cette seconde vague épidémique, la situation d'isolement ou de quarantaine n'est plus visée par la nouvelle

L'analyse juridique de la Caisse de prévoyance sociale démontre qu'elle ne disposerait pas des outils juridiques légaux pour répondre à cette situation. Elle reste toutefois dans l'attente de consignes nationales qui permettraient de débloquer la situation. À ce titre, je souhaite que le Gouvernement réactive le dispositif d'arrêt de travail dérogatoire pour toute personne placée en quarantaine ou à l'isolement à son arrivée en outre-mer et pour qui le télétravail est impossible. Ma demande vaut pour Saint-Pierre-et-Miquelon, mais également pour l'ensemble de l'outre-mer.

Je pense en particulier aux spécificités insulaires. La situation de Saint-Pierre et Miquelon appelle donc toute notre attention. C'est pourquoi une disposition réglementaire a été prise pour permettre de couvrir l'isolement des assurés sociaux arrivant sur l'île par des indemnités dérogatoires, afin notamment qu'ils ne soient pas concernés par le délai de carence. Par ailleurs, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon s'est attaché à identifier les besoins pour assurer un dispositif de septaine qui réponde à cet impératif de protection, mais qui soit aussi pleinement opérationnel. Ce travail a été mené en concertation avec la Caisse de prévoyance sociale, de manière à adapter le dispositif national à cette situation particulière. C'est à la suite de son alerte

sans délai de carence, dès leur arrivée sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et leur mise en septaine. Soyez donc assuré, monsieur le sénateur, que le Gouvernement est pleinement mobilisé pour que nos réponses à la crise sanitaire soient bien en phase avec la spécificité des territoires.

Les essais cliniques sont achevés et les résultats sont éloquents, avec une sensibilité de 88 % et une spécificité de 99,4 %, largement plus élevées que pour les tests antigéniques. quatre atouts majeurs : une grande simplicité de mise en oeuvre sur le terrain, grâce à un appareil nomade appelé « EasyVID », lequel permet de mailler très rapidement le territoire en traitant les sites prioritaires, comme les Ehpad ; un délai d'obtention des résultats de quarante minutes ; un coût très faible ; une démarche 100 % française, de la recherche à la production du système, en Vendée, par la société Tronico-Alcen. Je précise que ce programme est soutenu par la direction générale de l'armement et l'Agence de l'innovation de défense. Dans l'attente de l'homologation en France, des évaluations sont en cours dans 16 Ehpad de la Vendée, sur l'initiative unique du département. Le système est exporté aujourd'hui, mais ne peut être généralisé dans notre pays. Aussi, madame la ministre, pouvez-vous nous assurer que tout sera mis en oeuvre pour obtenir en urgence son homologation par la Haute Autorité de santé ?

vous m'interrogez sur le déploiement de nouveaux tests de dépistage de la covid-19, en particulier le test EasyCOV, développé par l'entreprise vendéenne Tronico. Il s'agit d'un test de type RT-LAMP, technique d'amplification génique proche de la RT-PCR. EasyCOV puise spécifiquement sur des prélèvements salivaires. La Haute Autorité de santé a validé l'utilisation de tests d'amplification génique sur prélèvement nasopharyngé le 6 mars dernier. Ces tests sont pris en charge à 100 % par la sécurité sociale depuis le 28 mai. La RT-LAMP est une technique déjà employée aujourd'hui dans des laboratoires d'analyses médicales. En ce qui concerne les prélèvements salivaires, la Haute Autorité de santé a, à ce jour, validé son utilisation uniquement pour la RT-PCR chez les patients symptomatiques. L'inscription sur la plateforme ministérielle des tests d'amplification génique, comme les tests EasyCOV, s'appuie sur deux critères non cumulatifs ils doivent soit disposer d'un marquage CE, avec une déclaration préalable à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, soit disposer d'une évaluation favorable de leurs performances par le Centre national de référence des virus des infections respiratoires. Le ministère n'a reçu aucun élément de ces deux institutions pour l'inscription du test EasyCOV. À ce stade, des échanges ont lieu avec les chercheurs autour de la question des tests salivaires pour pouvoir en démontrer la fiabilité dans le diagnostic virologique. Des évaluations complémentaires sont en cours concernant l'utilisation de ces prélèvements. Cette technique intéressante est suivie de très près. Je peux vous assurer, monsieur le sénateur, que le ministre des solidarités et de la santé est pleinement mobilisé pour mettre en valeur le savoir-faire de nos entreprises et s'assurer que nous disposons de tous les outils nécessaires

très bureaucratique- il faut le dire -, nous prive de résultats rapides en matière de tests salivaires. Je répète que ce système a été déployé dans un grand nombre de pays dans le monde ; la France, qui le produit à 100 %, n'est pas capable de le prendre en compte à très court terme.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, la direction de Bridgestone a annoncé, jeudi dernier, la fermeture de son site de Béthune, plongeant dans la colère et le désarroi les 863 salariés de cette entreprise. Mme la ministre chargée de l'industrie, que je côtoie régulièrement à la table des négociations, le sait bien : aucune des options permettant de continuer l'activité n'a trouvé grâce aux yeux de la direction du groupe, qui, pendant toute cette période, a joué la montre, manifestant le plus grand mépris à l'égard des salariés, des sous-traitants et de leur famille. Il est désormais évident que la fermeture de l'usine était cyniquement programmée depuis des années, faute d'investissements. Seule comptait la rentabilité du groupe Bridgestone, parfaite illustration de la logique destructrice du libéralisme. Sur le terrain, les territoires et leurs élus, les régions, les départements, les agglomérations se mobilisent et font preuve d'inventivité pour panser les plaies de l'exode de nos entreprises. Mais nous ne pouvons que constater l'absence d'une politique industrielle nationale solide, l'impuissance de l'Europe à nous protéger et l'incapacité de la France à faire bouger les lignes scénario, qui s'est trop souvent reproduit dans notre pays au nom d'une mondialisation dite « heureuse », ce sont les salariés de Bridgestone, après tant d'autres, qui le subissent

ni contreparties ? Quand allez-vous tirer les leçons de ces échecs et donner enfin à la France les moyens de reconquérir cette souveraineté industrielle que les territoires ont tant besoin d'offrir à ceux qui travaillent et créent la richesse de notre pays ? La parole

je sais combien vous êtes impliquée, comme votre collègue qui vient de poser une question sur le même sujet, aux côtés des élus du territoire, aux côtés de l'intersyndicale, aux côtés de la région et de l'agglomération, pour trouver une solution pour ces 863 hommes et femmes,

Aujourd'hui, il me semble que nous pouvons avancer justement grâce aux outils du plan de relance et à l'implication des élus du territoire et de l'intersyndicale,

et nous avons dit très directement à la direction de Bridgestone que le compte n'y était pas sur le plan social- vous connaissez l'implication de ma collègue Élisabeth Borne et de ses équipes sur ce sujet. Nous examinons de très près ce qui est proposé et nous aurons un observateur dans les négociations à venir à partir de demain. S'agissant des possibilités de reprise, non seulement nous avons mis la pression sur Bridgestone pour trouver des solutions des solutions de reprise, mais nous travaillons également avec Business France et avec l'ensemble des équipes de l'État, de la région et de l'agglomération pour contacter nous-mêmes des repreneurs potentiels.

Étudiants, jeunes, familles monoparentales, artisans, commerçants, extras, intérimaires, autoentrepreneurs, salariés fragilisés par le chômage partiel, voilà les nouveaux profils de ceux qui, aujourd'hui, basculent dans la précarité,

Comment rester imperméable à un drame pareil ? Les mois se suivent et apportent leur lot de statistiques effrayantes. L'aide alimentaire est l'un des thermomètres qui affichent les résultats les plus frappants : 8 millions de personnes en France n'arrivent plus à se nourrir. Les associations constatent une hausse de 25 % des demandes d'aide alimentaire.

Nous ne pouvons pas détourner le regard. Il faut désormais nous prémunir contre un autre mal, l'indifférence face à la vulnérabilité de nos plus fragiles. Monsieur le Premier ministre, les sénateurs de notre groupe ont fait de nombreuses propositions pour leur venir en aide réellement et le plus rapidement possible. Les réponses à l'urgence sociale ne peuvent souffrir aucun clivage politique. Pourtant, nous n'avons guère été entendus jusqu'à présent. J'espère que ma question en sera l'occasion ! Le but de celle-ci n'est pas de vous entendre dresser la liste des actions temporaires mises en place au printemps dernier- nous les connaissons -, mais je n'aurai de cesse de vous alerter sur l'urgence d'intensifier notre combat contre la pauvreté de nos concitoyens. Pouvez-vous nous dire clairement si le « quoi qu'il en coûte » s'adresse aussi à ces nouveaux visages de la précarité ? Ils sont 9,3 millions à ce jour. Combien seront-ils demain ? La pauvreté ne disparaît pas avec le virus, monsieur le Premier ministre : au contraire, elle ne fait que commencer

comme vous le soulignez, la situation sanitaire, économique et sociale est bien évidemment dramatique pour nos compatriotes les plus vulnérables. La pauvreté, comme vous le dites, n'est pas morte avec le covid, mais elle n'est pas non plus née avec attendu la crise sanitaire pour apporter des réponses aux besoins des Françaises et des Français, notre politique de solidarité à destination de nos concitoyens a été renforcée pour permettre à chacune et chacun de surmonter la situation.

pour l'accès aux soins optiques, dentaires et auditifs, qui sont intégralement pris en charge par la solidarité nationale. Le Ségur de la santé consacre 100 millions d'euros par par an à la lutte contre les inégalités de santé. Nous protégeons les plus fragiles, avec la reconduction automatique des minima sociaux et près de 3 milliards d'euros d'aides directes à nos concitoyens.

Enfin, ce sont 100 milliards d'euros qui sont mobilisés dans le plan de relance pour permettre à notre économie de tenir le choc et d'assurer une relance créant des emplois pour nos concitoyens, en particulier pour les jeunes. 6,5 milliards d'euros qui sont mobilisés dans le plan « 1 jeune, 1 solution », pour la formation, l'insertion et l'embauche de plusieurs centaines de millions de jeunes. Vous l'aurez compris, madame la sénatrice, la sénatrice, nous agissons concrètement pour apporter une réponse d'ensemble et, ainsi, permettre à nos concitoyens de faire face aux conséquences de cette crise sociale majeure, qui dure. Le Gouvernement veillera activement à ce qu'aucun de nos compatriotes en difficulté ne soit laissé sur le bord du chemin. La parole

Le Jura est le pays du jouet et Moirans-en-Montagne, sa capitale. C'est le siège de Smoby, premier fabricant français de jouets, mais aussi de nos autres créateurs de merveilles : Vilac, Janod, Juratoys, Jeujura, Roz, Charliluce, etc. 60 % du chiffre d'affaires se fait en deux mois, 70 % dans les magasins spécialisés ou en grandes surfaces. Le ne suffira pas à compenser les pertes causées par la fermeture des boutiques. Pis, le spectre du Black Friday vient tourmenter l'ensemble des commerçants. Avec 6 milliards dépensés en 2019, c'est un week-end qui compte triple, comme le souligne Bruno Le Maire. Avec une réouverture des commerces programmée le 1 décembre, le Black Friday, le 27 novembre, est plus qu'une provocation : c'est une mise à mort. Monsieur le Premier ministre, il fallait bien le reconfinement pour casser la nouvelle vague épidémique. Mon département, le premier, en avait grand besoin. Vous avez réussi à enrayer la progression du virus et ses conséquences si dramatiques. Mais force est de constater qu'aujourd'hui la covid-19 prive d'oxygène et ses victimes, et notre système économique tout entier, pour lequel il n'y aura pas de vaccin. Le pic épidémique est passé. C'est maintenant à Olivier Véran de veiller sur Bruno Le Maire ... Monsieur le Premier ministre, vendredi 27 novembre, cela fera exactement quatre semaines que les Français auront consenti à tous les efforts que vous jugiez nécessaires, quatre semaines que nos commerçants cherchent à survivre. Peuvent-ils vous demander un effort de quatre jours ? La

à qui je veux rendre un hommage appuyé. Comme vous le savez, j'ai reçu, il y a une dizaine de jours, Smoby et tous les fabricants de jouets en bois du Jura qui perpétuent une tradition séculaire de fabrication de jouets dans votre département. Je sais, comme chacun d'entre vous ici, à quel point la situation est difficile pour eux, qui font 60 % à 70 % de leur chiffre d'affaires dans les dernières semaines précédant Noël. Ils n'attendent qu'une seule chose : pouvoir rouvrir et vendre leurs jouets. Croyez-moi, avec le Premier ministre et le Président de la République, nous faisons le maximum

dates. J'ai toujours rappelé, dans cet hémicycle et ailleurs, que nous ne gagnerons la bataille contre le virus et la bataille économique que si chacun fait preuve de sens des responsabilités.

et d'examiner toutes les possibilités de décaler cette opération, qui n'a pas de sens dans les circonstances actuelles. La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour le groupe Les Républicains. Ma question

le vendredi 6 novembre, lors de la réunion du comité stratégique de la filière automobile, vous avez demandé la prolongation pour six mois des aides à l'achat de voitures neuves, à l'exception des voitures hybrides diesel, qui seront exclues du dispositif à compter du 1 janvier 2021. Ce faisant, vous avez officialisé ce que beaucoup redoutaient depuis la déclaration de Mme la ministre de la transition écologique sur Twitter le 12 octobre dernier : vous avez fait le choix de condamner le diesel hybride. Vous avez fait ce choix sans attendre les résultats de l'étude scientifique indépendante, pourtant sollicitée par le Gouvernement en 2019, lorsque vous vous disiez favorable à ce que les nouveaux véhicules diesel moins polluants puissent être éligibles à la vignette CRIT'Air Cette politique économique conduit à aggraver la désindustrialisation de la France dans de nombreux territoires, alors même que le Président de la République appelle à relocaliser l'industrie sur le sol français. Les discours sur la réconciliation entre industrie et écologie ne trompent personne lorsqu'ils nous sont démentis par les faits. Bien évidemment, le diesel de seconde génération doit prendre part à la transition écologique, mais, par vos mesures, vous faites un autre choix et les usines ferment. Concrètement, en Aveyron, l'usine de l'équipementier allemand Bosch d'Onet-le-Château, plus gros employeur du bassin d'emploi de Rodez, est menacée par la suppression d'au moins 30 % des emplois du site et plus encore par l'éventualité d'une fermeture définitive, évoquée lors du dernier comité social économique de l'entreprise. Aussi, monsieur le ministre, pourquoi condamner définitivement la filière automobiles diesel en France, dont les efforts, dans le cadre de la transition écologique, sont considérables et alors que vous sembliez la soutenir voilà encore six mois ? Que comptez-vous faire pour sauver le site aveyronnais Bosch d'Onet-le-Château ? Pourquoi faire le choix de Pourquoi faire le choix de la désindustrialisation et du sacrifice de milliers d'emplois au profit d'une transition écologique mal appliquée ?

en dépit des campagnes de communication menées par le royaume, l'Arabie saoudite continue les détentions arbitraires des militants des droits de l'homme : l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, par exemple, reste impuni à ce jour.

! Emprisonnée sans perspective de procès équitable, elle fait aujourd'hui la grève de la faim. D'autres femmes sont torturées à l'électricité ou à coups de fouet ou subissent des sévices sexuels pour avoir demandé la fin du système patriarcal. Toutes sont réprimées

tout simplement. La France ne peut tolérer cela ! Dans ce contexte de violations répétées des droits de l'homme en Arabie saoudite, quelle sera la position de la France lors du G20 ? Vous n'en avez, à ce jour, pris aucune. Or le G20 est Or le G20 est l'occasion de montrer au monde que la France est toujours capable de défendre les libertés fondamentales. Monsieur le secrétaire d'État, allez-vous prendre vos responsabilités et mettre l'Arabie saoudite devant les siennes ?

Tous les conseils de sécurité se sont réunis ou vont se réunir. Nous portons la plus grande attention à renforcer les dispositifs aux abords de nos écoles, en lien avec les autorités locales. Ce n'est

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie. Madame la ministre, en octobre 2019, le Gouvernement a présenté un plan de mobilisation nationale pour l'attractivité des métiers du grand âge.

Cette prime, dénommée « grand âge », est de nature pérenne et vise à reconnaître l'engagement et les compétences professionnelles des aides-soignants, mais aussi à motiver les candidats en revalorisant leur statut et leur salaire. Madame la ministre, les remontées du terrain font pourtant apparaître des inégalités de traitement selon les structures dans lesquelles travaillent les aides-soignants

il est impossible de demander à nos communes, à nos maires, à nos collègues de financer cette nouvelle dépense alors que les dotations de l'État ne cessent de diminuer. ! Finalement, au lieu d'améliorer les choses, le Gouvernement crée un déséquilibre de traitement qui aggrave les difficultés de recrutement de nos maisons de retraite gérées par nos communes, par nos centres communaux d'action sociale, par les associations ou par les fondations, au profit des Ehpad hospitaliers.

Le plan Hôpital présenté voilà un an par Agnès Buzyn était la première brique d'un investissement de l'État en faveur de la revalorisation de ces métiers. Comme vous le savez, ce plan prévoyait la création d'une prime « grand âge » à destination des infirmiers, des aides-soignants et des aides médico-psycho dans les Ehpad publics. Cette prime est

si les partenaires sociaux souhaitaient la mettre en place. Ce point est donc laissé à leur appréciation, dans le respect de leur liberté de négociation. À ce jour, aucun accord en ce sens n'a été conclu, et les financements associés n'ont donc pas été délégués. Voilà quelle La balle est dans le camp des partenaires sociaux. Je veux le rappeler, à cette revalorisation de la prime « grand âge » s'ajoute celle que les accords de Ségur à hauteur de 183 euros par mois, pour les Ehpad publics et privés non lucratifs et de 160 euros par mois pour les Ehpad privés commerciaux. Cette mesure vaut pour tous les personnels de tous les Ehpad. Elle est entièrement financée par la branche autonomie,

Depuis le début de la crise, les fédérations du sport amateur ont perdu en moyenne entre 10 % et 30 % de leurs licenciés et des centaines de millions d'euros de recettes, qui ne manquera pas d'avoir des conséquences sur l'activité économique de nos territoires et sur le lien social- n'oublions pas que le sport est l'un des moyens pour nos jeunes d'échapper aux addictions et à la délinquance. Le sport professionnel est tout aussi durement touché. En qualité de président de l'amicale parlementaire du rugby, au nom de mes 120 collègues membres, je voudrais vous dire combien la situation est difficile dans notre sport, qui dispose, avec le Top 14, du meilleur championnat au monde. À trois ans de l'événement majeur qu'est la Coupe du monde de rugby France 2023, nos clubs risquent de se retrouver singulièrement menacés, et l'équipe de France, malgré ses derniers résultats encourageants, singulièrement affectée.

sont, comme le rugby, menacés dans leur existence même, car leurs recettes dépendent essentiellement des spectateurs et des hospitalités. Monsieur le Premier ministre, si 2 milliards d'euros ont été versés pour venir en aide à la culture, ce dont nous nous félicitons, pouvez-vous nous détailler les 400 millions d'euros qui concernent le sport, professionnel ou amateur, qui joue un rôle si essentiel dans notre société ?

que les clubs, les maisons sport-santé et les salles de sport aient un minimum d'activité pour garder intact ce lien de confiance qu'ils ont mis des années à tisser avec leurs adhérents. J'ai donc insisté, hier, pour que l'activité sportive des mineurs puisse reprendre dans les clubs dès le mois de décembre prochain, avec des protocoles sanitaires renforcés,

La séance est reprise. Mes chers collègues, les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat. En l'absence d'observations, je les considère comme adoptées.-

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, deux ans après l'examen en première lecture de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, ou ANCT, et près d'un an après sa création juridique, le groupe RDSE a tenu à faire un point sur l'évolution de la mise en place de cette structure, non pas pour établir un bilan exhaustif de son action, mais pour permettre à l'ensemble des groupes parlementaires du Sénat- la chambre des territoires -, de s'exprimer sur leurs attentes légitimes.

Cette carence accentue la fracture territoriale, creusée par des années de déclin de la politique de l'aménagement du territoire, par le retrait de l'État stratège. Elle a eu pour conséquence d'accentuer la concurrence entre les territoires, plutôt que de favoriser leur solidarité. Au-delà des enjeux relatifs à la transformation de l'économie et de l'emploi, aux mobilités et à l'accès aux services publics, notre pays doit s'engager résolument vers la transition écologique, énergétique et numérique de ces territoires, en révélant leur potentiel. Les bénéfices de cette charge collective et de ces opportunités doivent profiter à tous, en tout point du territoire. La crise sanitaire conforte la volonté des élus locaux d'accroître la résilience économique, mais aussi durable, de nos territoires, garante d'une relance pérenne. Que demandent les élus ? De l'équité, les mêmes chances de développement pour tous et un rééquilibrage des forces économiques permettant d'adapter le maillage de nos services publics, donc de répondre aux besoins de nos concitoyens. Rien de plus, rien de moins, sinon la stricte déclinaison de l'article I de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». l'État doit soutenir l'autonomie des collectivités territoriales et intervenir là où c'est strictement nécessaire. L'ingénierie administrative, juridique et financière constitue un instrument fondamental là où l'initiative privée ou publique n'a pu se déployer.

transformer l'action publique déconcentrée au plus près de nos concitoyens et passer d'un État Léviathan à un État protecteur et facilitateur, qui, en renforçant l'efficacité de la déconcentration, vient soutenir l'exercice de la décentralisation. Nos concitoyens et les élus qui portent leurs aspirations n'ont pas besoin de contraintes normatives supplémentaires, ni d'une nouvelle structure se plaçant au-dessus de l'existant, ni d'un ralentissement de la prise de décision. Nous ne voulons ni plus d'État ni moins d'État. Nous voulons mieux d'État, accompagnement des élus portant des projets indispensables pour la vitalité de leur territoire, qui sont parfois freinés par un excès de bureaucratie tatillonne. Le deuxième élément du diagnostic était la complexité administrative. À défaut de réussir la simplification des normes ou des circuits de financement, nous espérions proposer aux collectivités locales un accès aisé à leur application ou à leur recours, grâce à une logique de guichet unique. de guichet unique. Tel était l'objet premier de l'ANCT, tel que nous l'envisagions. Il s'agissait de rompre avec les répercussions négatives sur les collectivités de la verticalité et du cloisonnement des services administratifs. Cela supposait de doter l'administration territoriale des moyens correspondants, alors que les effectifs des directions départementales des territoires et de la mer, les DDTM, ont subi une perte de 30 % de leurs effectifs entre 2012 et 2018 et rencontrent actuellement des difficultés à assurer l'ensemble de leurs missions. Force est de le constater, ces moyens n'augmenteront pas en 2021, malgré l'accroissement de la charge de travail des préfectures, lesquelles ne cessent d'être sollicitées depuis la crise sanitaire. Le rapport d'information portant sur l'ingénierie territoriale, remis en juillet dernier par Charles Guené et notre ancienne collègue Josiane Costes, recommandait la construction de ce guichet unique, « dans une culture de qualité de service et de résultat en confortant les moyens des services déconcentrés de l'État [ ...] et en association avec ses partenaires locaux ». Par ailleurs, il s'agissait de sortir de la logique des appels à projets.

auxquels les territoires répondaient. Bien évidemment, je n'ai pas besoin de vous rappeler que, de manière générale, c'étaient toujours les mêmes territoires qui répondaient à ces appels, à savoir ceux qui disposaient de moyens techniques et financiers. Sans contester l'utilité des programmes nationaux, il n'y a pas eu d'inflexion quant au recours aux appels à projets, et nous nous interrogeons quant à la place qui restera pour les projets émanant des collectivités. C'est le service sur-mesure que nous espérions voir renforcé. À ce titre, le groupe RDSE avait fait adopter un amendement visant à doubler l'enveloppe consacrée à l'ingénierie territoriale, lors de l'examen de la loi de finances pour 2020. Ce doublement est repris dans le projet de loi de finances pour 2021, et nous nous en réjouissons de ce premier pas. Enfin, l'administration doit se réformer et faire cohésion. C'est le sens du recours à une agence, puisque, conformément à la définition retenue par le Conseil d'État, elle n'est ni indépendante ni inscrite dans le schéma traditionnel de l'administration centrale et de ses services déconcentrés.

L'instauration d'un guichet unique suppose donc un changement de culture administrative. Certes, la transformation de l'action publique ne peut se faire en un an, encore moins dans un contexte de crise. Il ne serait pas juste de dresser un bilan prématuré, mais il est temps d'engager un changement de modèle et de travailler en mode projet, comme le recommandait Serge Morvan, dans son rapport de préfiguration de l'agence. Mes chers collègues, monsieur le secrétaire d'État, nous ne sommes pas en guerre, bien que certains puissent affirmer le contraire. Cependant, en guise

Les services du département de la guerre ne sont pas tous suffisamment dégagés de certaines méthodes de travail, dont la lenteur ne correspond pas aux nécessités de l'heure présente. Les errements du temps de paix continuent. Il est urgent qu'une chasse obstinée soit faite à tous les temps morts qui ralentissent encore la machine administrative : l'intérêt du pays l'exige. » La parole est à M. le

Certes, contrairement à ce qu'indique l'intitulé du débat, l'ANCT n'a pas tout à fait un an, puisqu'elle a été créée le 1 janvier 2020. Par ailleurs, si l'agence a bien été juridiquement créée en janvier 2020, la fusion des personnels, l'élaboration de l'organigramme et celle de sa feuille de route, ainsi que les négociations en vue de la signature des conventions pluriannuelles avec d'autres opérateurs ont nécessité plusieurs mois de travail. Il est donc temps, à l'approche de ce premier anniversaire, de dresser un premier bilan de ce jeune établissement public. Je voudrais d'emblée, avant de répondre à vos questions, remercier les services de l'ANCT de leur concours indispensable et efficace, dont je me rends compte quotidiennement en ma qualité de secrétaire d'État à la ruralité. Les services de l'ANCT ont été mis à disposition de mon ministère, dans le cadre de la politique de développement des territoires ruraux, qui m'a été confiée par le Président de la République et le Premier ministre. À ce titre je suis notamment chargé du suivi de la mise en oeuvre de l'agenda rural, une politique dont l'ANCT assure la coordination. Les avancées du dernier comité interministériel, qui s'est tenu le 14 novembre dernier, ont été saluées de toutes parts. Elles montrent tout l'apport de l'ANCT dans le travail interministériel et l'intérêt d'avoir un opérateur spécialisé. À cette occasion, nous avons engagé un nouveau dispositif prévu par l'agenda rural, auquel je tenais beaucoup, à savoir le volontariat territorial en administration, le VTA, sur le modèle du VTE, le volontariat territorial en entreprise. Ce dispositif est de nature à renforcer l'ingénierie à disposition des territoires et des petites collectivités. En effet, ce sont, à terme, 800 jeunes qui pourront bénéficier de cette possibilité, donc 800 collectivités qui seront accompagnées en ingénierie, notamment dans le temps du plan de relance. Les jeunes VTA apporteront un concours précieux à ces collectivités pour monter leur projet. En retour, ils acquerront une expérience professionnelle valorisante. C'est que j'appelle du gagnant-gagnant, au service des territoires et de la jeunesse. Nous montons également, dans le cadre de l'agenda rural, des partenariats renforcés avec certains ministères, pour enrichir le soutien que nous apportons aux collectivités locales. C'est le cas pour le déploiement des projets alimentaires territoriaux. En lien avec le ministère de l'agriculture, 80 millions d'euros ont été ouverts, dont 5 millions d'euros en ingénierie. Comme vous le constatez au travers des avancées du comité interministériel aux ruralités, le Gouvernement partage votre point de vue sur l'importance de l'ingénierie dans les territoires. Il fait donc en sorte que l'ANCT complète son offre en la matière. L'ANCT a également pour objectif de simplifier la relation entre les élus locaux et l'État. le rappelle, la création de l'agence visait à répondre au souhait exprimé par les élus locaux de disposer d'un accès simple aux services de l'État et aux différents opérateurs qui interviennent pour soutenir leurs projets. L'organisation de l'ANCT est d'ailleurs déconcentrée, et les préfets sont les délégués départementaux de l'ANCT dans les territoires. Les commissariats de massifs sont également des relais territoriaux de l'agence dans les massifs de montagnes. Les associations d'élus participent directement au conseil d'administration de l'agence, qui est présidé par Caroline Cayeux, la maire de la ville de Beauvais. En outre, au travers de ses divers programmes nationaux d'intervention, l'agence est aussi le bras armé de la politique de cohésion des territoires. J'ai cité l'agenda rural et l'organisation récente du comité interministériel. Nous avons également lancé la conception d'un programme dédié à la montagne, lors du congrès de l'ANEM, l'Association nationale des élus de la montagne, qui devrait aboutir à la mi-mai 2021.

Le programme Petites villes de demain a été lancé le 1 octobre 2020. Le comité interministériel aux ruralités a été l'occasion d'annoncer la première vague de labellisations, avec 170 communes sélectionnées dans trois régions : PACA, ou plutôt Sud,

Pour cette ingénierie sur mesure, une enveloppe de 20 millions d'euros, soit 10 millions supplémentaires par rapport à 2020, est prévue dans le projet de loi de finances pour 2021, comme vous l'avez souligné, monsieur Requier. Le doublement des crédits d'ingénierie de l'ANCT constituait une demande forte du ministère dans le cadre des négociations budgétaires. En effet, bien souvent, ce ne sont pas les financements et les idées qui manquent ; c'est l'ingénierie qui fait défaut pour les plus petites collectivités. Notre objectif est de les aider à monter leurs projets et à se saisir des crédits que l'État met à leur disposition. Je pense en particulier aux crédits de la relance, pour le déploiement desquels nous comptons énormément sur les territoires. À cette fin, l'ANCT sera pleinement mobilisée pour assurer la déclinaison et la réussite du plan France Relance. La philosophie de ce plan, vous le savez, est une réponse territorialisée à la crise. Je partage avec le Premier ministre la conviction que la relance se fera par les territoires. C'est pourquoi nous avons opté pour une large déconcentration des crédits au niveau des préfets. L'ANCT a participé aux travaux préparatoires du plan de relance et a contribué à nourrir la réflexion gouvernementale dès le printemps et durant tout l'été. C'est ainsi que plusieurs chapitres du plan de relance concernent directement ou indirectement l'ANCT. Outre la mobilisation exceptionnelle de 250 millions d'euros sur deux ans du Fonds national d'aménagement et développement du territoire, le FNADT, outre les programmes nationaux que j'ai cités et qui se voient allouer de nouveaux moyens, l'ANCT assurera la gestion du fonds de subventions d'investissement mis en place par l'État, pour soutenir les opérations de restructuration des locaux d'activité dans le cadre de création de foncières de redynamisation territoriale. Ce fonds représente 180 millions d'euros, dont 60 millions sur les deux premières années. L'ANCT est également mobilisée sur plusieurs autres volets du plan de relance, comme la rénovation énergétique des bâtiments, l'inclusion numérique, avec la généralisation de la fibre d'ici à 2025 et les opérations de rénovation des réseaux électriques, d'eau potable ou d'assainissement. Pour résumer, l'ANCT, je tiens à le souligner, sera présente dans l'ensemble du champ de l'action publique : industrie, transition écologique, mobilité, jeunesse, numérique et culture. Forte de son expérience en matière de contractualisation avec les collectivités, l'agence sera impliquée dans l'élaboration des contrats de relance et de transition écologique, qui prendront la dénomination de contrats de ruralité de transition écologique dans les territoires ruraux, qui permettra une diffusion rapide de ces contrats sur les territoires. En conclusion, madame la présidente, monsieur Requier, mesdames, messieurs les sénateurs, l'agence est désormais pleinement opérationnelle et répond aux objectifs que lui avait fixés la loi du 22 juillet 2019. Nous allons débat interactif. Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

Les collectivités territoriales ont dû faire face ces derniers mois à la crise de la Covid. Le déploiement des projets a dû s'effacer temporairement face à l'urgence sanitaire. Les dégâts de la crise actuelle mèneront sans doute à une sollicitation accrue des collectivités, qui souhaiteront les réparer et assurer, par exemple, une revitalisation de leur centre-ville,

à renforcer le besoin d'individualisation de l'accompagnement pour la mise en place de nouvelles ambitions de gestion et de soutien pour la mise en oeuvre de projets de territoire, plus durables, afin de faire face à des défis tels que la transition énergétique. Si l'ambition première de l'ANCT est l'ingénierie d'appui, que ce soit d'un point de vue réglementaire, juridique, financier, administratif ou de projets, plusieurs points restent encore sans réponse. Ils concernent l'efficacité réelle ou espérée du dispositif et sa capacité à répondre à la demande de recherche d'équilibre et d'équité entre les territoires. J'en pointerai deux, avec une bienveillance naturelle pour un nouveau-né que nous espérons voir se développer harmonieusement et rapidement. Premièrement, l'agence se veut l'outil de simplification des démarches. Je souhaiterais connaître les modalités d'évaluation de l'impact que l'ANCP pense apporter. Comment allez-vous évaluer l'efficacité de cet outil en termes de services rendus aux collectivités ? Gain de temps ? Baisse des coûts des projets ? ... Deuxièmement, les collectivités territoriales sont parfois enracinées dans un tel qu'elles cherchent toujours un appui auprès de certains organismes.

Par ailleurs, la présidence du conseil d'administration est confiée à une élue, qui est la présidente de Villes de France et qui me semble particulièrement efficace sur le terrain. Au niveau local, des comités locaux de cohésion territoriale sont présidés par le préfet de département,

Buis. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier le groupe RDSE de ce débat important, qui se tient quasiment un an après la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Monsieur le secrétaire d'État, l'une des principales missions de l'Agence nationale de la cohésion des territoires est d'accompagner les projets des collectivités les plus fragiles, que celles-ci soient urbaines, périurbaines, rurales ou ultramarines, en prenant en compte leurs spécificités territoriales. L'État doit être facilitateur pour les collectivités. À cet effet, l'agence disposait pour l'année 2020 d'un soutien à hauteur de 54 millions d'euros au titre de sa subvention pour charges de service public. Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit une augmentation de 7 millions d'euros, portant ainsi ce montant à 61 millions d'euros, afin de permettre le doublement du montant de l'ingénierie destinée à appuyer des projets sur mesure, portés par les territoires. Avec une telle augmentation de son budget, plus de 300 équivalents temps plein à disposition, et un contexte sanitaire accentuant la fragilité des territoires, comment l'ANCP entend-elle participer à la mise en oeuvre du plan de relance dans ces territoires ? En effet, son engagement auprès des territoires les plus fragiles, au même titre que la mobilisation de l'ensemble des acteurs ruraux, est impératif pour relever les défis de la relance. La parole

à la crise, s'appuyant sur les territoires, qu'il s'agisse des collectivités territoriales ou des services déconcentrés de l'État, est en parfaite concordance avec les démarches poursuivies par l'agence.

l'agenda rural, ou encore à tous les programmes de la politique de la ville, qui pourront s'appuyer sur des crédits ouverts au type des différentes actions qui sont conduites par le plan de relance. Ainsi, pour ce qui concerne le programme Territoires d'industrie, piloté en lien avec le ministère chargé de l'industrie et les régions, un fonds de 400 millions d'euros sur la période 2020-2022, dont 150 millions d'euros dès 2020, est créé dans le cadre du plan de relance, pour soutenir les projets d'investissements industriels dans ces territoires. Par ailleurs, forte de son expérience en matière de contractualisation avec les collectivités, l'ANCT sera pleinement impliquée dans le pilotage et la coordination des contrats territoriaux de relance et de transition écologique. La contractualisation avec les collectivités territoriales participera pleinement à la réussite de ce plan de relance. Cela permettra d'associer les collectivités au financement des actions, afin de créer un effet de levier sur les crédits de l'État. Enfin, nous aurons l'occasion d'évoquer ce point à plusieurs reprises au cours du débat, l'accompagnement sur mesure des projets optimisera la mobilisation de l'ingénierie nécessaire à la réalisation effective des opérations. Les crédits supplémentaires du plan de relance permettront de répondre massivement et rapidement aux saisines des collectivités qui souhaitent

Les missions qui lui ont été confiées en termes de conseil et de soutien aux collectivités dans la mise en oeuvre de leurs projets la rendront, je l'espère, incontournable auprès des territoires, notamment les territoires hyper-ruraux, comme mon département de la Lozère.

Ainsi, nombre de territoires en manque de moyens financiers ne peuvent répondre aux appels à projets, ce qui alimente la concurrence entre territoires, au profit des pôles urbains. la demande d'ingénierie, en proposant de faire de l'ANCT le pivot de la mutualisation et des ressources locales. Les propositions 15 et 16 de ce rapport prévoient notamment la création d'une plateforme numérique centralisant les moyens d'ingénierie publique et la diffusion des bonnes pratiques, par un retour d'expérience sur l'espace « projet ». Cette notion de diffusion et de partage est, selon moi, centrale si l'on souhaite non pas alimenter la concurrence, mais bien faire primer l'alliance entre nos territoires.

Vous avez raison de le souligner, cette notion de diffusion et de partage est primordiale, notamment grâce à la centralisation des moyens d'ingénierie publique et la diffusion des bonnes pratiques par un retour d'expérience sur l'espace « projet La loi créant l'ANCT a donné à cette dernière la mission de « faciliter l'accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d'ingénierie juridique, financière et technique qu'elle recense [ ...]. » La disponibilité des ressources en ingénierie est aujourd'hui extrêmement morcelée et inégalement accessible sur le territoire. Les acteurs sont nombreux. Ils proposent des aides financières, des dispositifs

plateforme Aides-territoires, qui est développée dans le cadre de la Fabrique numérique par le ministère de la transition écologique. C'est un portail internet qui référence les aides, qu'elles soient ou non financières, à tous les territoires. Il s'adresse aux agents des collectivités

d'offrir à toutes les collectivités le même niveau d'information et de faciliter et d'améliorer la communication sur les aides publiques pour ceux qui les portent. Si vous y ajoutez les moyens locaux que nous allons mettre à disposition des collectivités- je pense en particulier aux VTA, les volontaires territoriaux en administration -, je pense que cette plateforme sera plus facile encore à manier avec le meccano qui se met en place.

monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il y a un an, le Parlement a donc voté la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, préfigurée par le rapport Morvan et censée incarner une vision profondément renouvelée de l'action de l'État dans les territoires. Cette structure a soulevé une vague d'espoir parmi les élus, qui en attendaient du soutien financier, mais également de l'expertise pour mener à bien leurs projets, surtout pour les plus petites collectivités. Celles-ci subissent en effet, et de plein fouet- nous en voyons beaucoup d'exemples dans nos départements ruraux -, l'affaiblissement de l'ingénierie des services de l'État sur le terrain et le désengagement, voire la fermeture, des services publics de proximité, ce recul se conjuguant avec une baisse continue des dotations. Pourtant, en cette période inédite, comment méconnaître qu'elles sont les acteurs incontournables de la relance ? Face à ce constat, malheureusement, l'agence peine toujours à convaincre. Tout d'abord, elle a confirmé nos craintes concernant un renforcement des pouvoirs des préfets, devenus omnipotents. Par ailleurs, au regard de l'ensemble de ses missions, son activité aura été bien faible et resserrée. Ainsi l'agence a-t-elle été sollicitée uniquement pour 81 projets, hors programmes nationaux ; sur ces 81 projets, 70 dossiers de restructuration commerciale étaient déjà en cours. D'autres dossiers relèvent d'une ingénierie sur mesure ; ceux-ci sont dotés d'une enveloppe doublée cette année à hauteur de 20 millions d'euros, une somme dérisoire. L'agence, qui devait également nouer des partenariats avec l'ensemble des acteurs de l'État pour la transition écologique, risque enfin d'être pénalisée par la perte de 800 postes parmi les opérateurs de l'État en matière d'écologie cette année. Quelle est donc la plus-value réelle de l'agence, dont la fonction essentielle est de jouer le rôle d'un guichet unique en mutualisant des moyens et des outils le plus souvent déjà existants, portés y compris par les départements ? Monsieur le secrétaire d'État, ma question sera simple : comment faire toujours plus avec toujours moins ? secrétaire d'État. Madame la sénatrice, je vous trouve un peu dure avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, tout simplement parce qu'il s'agit d'un nouveau-né, comme je l'ai dit ; et vous jetez déjà ce nouveau-né avec l'eau du bain ... Je ne pense pas que ce soit utile. Justement, si cette agence a été créée, c'est

Premièrement, comment éviterons-nous que l'agence soit simplement le bras armé de l'État pour aider des collectivités à répondre à des appels à projets qui sont souvent très frustrants et très mobilisateurs de temps ? Comment pourrait-elle devenir plutôt le bras armé des collectivités

les élus locaux puissent saisir, tout simplement, cette agence. Il y a, dans nos territoires, un vrai besoin d'ingénierie, non seulement en conception de projets mais aussi,

L'affaiblissement de l'État territorial a renforcé les inégalités en matière d'ingénierie et a contribué à ce sentiment d'abandon que, en tant qu'élus locaux, nous connaissons bien. L'ingénierie locale a souvent compensé efficacement ce retrait de l'État, mais de manière non uniforme. Les collectivités les plus fragiles, dépourvues d'équipes et de moyens suffisants, sont amenées à se focaliser sur une logique où les dépenses d'investissement, l'ingénierie opérationnelle notamment, l'emportent sur les études en amont, alors que celles-ci permettent justement d'économiser des moyens en aval. Face à cette situation, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est apparue comme le remède à la désertion de l'ingénierie publique d'État. En lieu et place du guichet unique annoncé et tant attendu par les élus locaux, l'ANCT serait une fabrique à projets à la main des préfets du département, apportant si elle le peut l'ingénierie nécessaire là où elle est défaillante. Ainsi, ce sont les territoires les plus vulnérables qui pourront bénéficier de l'ingénierie étatique, comme il est expliqué dans la feuille de route pour 2020 en date du 17 juin Pour le moment, l'ANCT est, pour les élus, une espérance davantage qu'une réalité concrète, mais une espérance tout de même. Le programme Petites villes de demain vient tout juste d'être lancé, les comités locaux s'organisent, des « contrats de relance et de développement écologique » ont été promis par le Premier ministre lors du deuxième comité interministériel aux ruralités qui s'est tenu samedi dernier. concrètement, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous préciser quelle complémentarité vous envisagez entre l'ingénierie locale et l'ingénierie nationale ? Va-t-il y avoir une contractualisation, une labellisation, une mutualisation ?

de cohésion territoriale ? Les comités régionaux des financeurs ? Voilà des questions simples, que se posent les élus et qui appellent des réponses simples. La le secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Bigot, vous m'interrogez essentiellement sur l'articulation concrète entre l'offre d'ingénierie proposée par l'ANCT et l'ingénierie locale. locale. Dans plusieurs départements, je le disais, ont été déployés des dispositifs d'ingénierie ou d'appui à l'ingénierie au profit des collectivités ; je pense par exemple à toutes les agences techniques départementales, mais aussi aux services, déjà en fonction dans plusieurs collectivités, qui réalisent ces missions dans des domaines parfois très larges. Cette dynamique d'ingénierie territoriale réaffirme notamment la place du département- vous avez en face de vous un membre du Gouvernement qui est plutôt départementaliste, parce qu'il est issu d'un territoire rural -dans son rôle d'assistance technique aux collectivités territoriales. L'offre de l'ANCT- je l'ai dit tout à l'heure à Mme Gatel, mais je le répète volontiers -n'a vraiment pas vocation à entrer en concurrence avec l'existant,

lorsqu'elles sont possibles- et elles sont possibles dans nombre de cas. Il faut s'assurer qu'une collectivité qui a un besoin auquel il peut aisément être répondu avec des moyens existants localement ne passe pas à côté faute d'en avoir eu connaissance ; en effet, cela arrive. Il s'agit aussi de permettre aux dispositifs existants d'être pleinement mis en oeuvre. Ainsi, je le répète, la complémentarité avec l'ingénierie locale est constamment recherchée : l'ANCT propose une offre de services d'ingénierie sur mesure, qui n'est activée que lorsque l'offre d'ingénierie disponible localement ne suffit pas. Elle est, en ce sens, particulièrement équitable : les départements qui n'ont pas été en mesure de mettre cette ingénierie en oeuvre pour des raisons par exemple financières

néanmoins saluer la présidente de l'agence, Caroline Cayeux, ainsi que son directeur général, Yves Le Breton, et toute son équipe, pour leur volonté de mettre en place un fonctionnement efficace et partagé fondé sur la coordination des opérateurs nationaux avec lesquels l'agence a contractualisé ainsi qu'avec les préfets de département.

Le doublement de ses crédits d'ingénierie pour 2021 est un signe positif ; j'espère que ce geste sera par la suite amplifié. Il faut avant tout éviter que les grandes agglomérations, mieux pourvues, aspirent l'essentiel des financements, au détriment des territoires les moins outillés, et arriver au « cousu main J'insisterai également sur l'importance des actions à mener pour garantir le rôle de l'agence et ses missions, en particulier auprès des territoires ruraux, dans la territorialisation du plan de relance. L'absence de toute référence à l'agence dans la circulaire du Premier ministre m'étonne et m'inquiète, alors que l'ANCT doit être l'outil des ministères sur les territoires. Enfin, concernant le guichet unique, je constate un réel risque de perte d'efficacité et de doublon entre les nouvelles instances du plan de relance et les comités existants de l'agence, ce qu'il faut absolument éviter. En conclusion, je forme le voeu que l'année 2021 montre l'efficacité de l'agence et clarifie le « qui fait quoi ». L'ANCT ne saurait être une simple réorganisation administrative d'agences de l'État sans moyens supplémentaires ; 2021 doit témoigner de sa performance dans la mise en place des politiques publiques au service des territoires,

acteurs locaux. La déconcentration est aussi extrêmement intéressante : elle permet un dialogue avec le préfet, délégué territorial officiel de l'agence, qui examine en premier ressort l'intégralité des sollicitations

L'année a aussi été marquée par l'installation de nouveaux élus locaux, qui devront faire face à la pandémie et à des reports d'élections. On voit les difficultés s'accroître et les demandes se diversifier. Nous ne devons pas oublier que l'objectif premier de l'ANCT est de favoriser et d'améliorer ce que l'on appelle communément l'ingénierie territoriale. Les mois et années qui viennent seront consacrés à la relance du pays. La territorialisation du plan de relance, que vous avez évoquée lors de votre audition il y a quinze jours par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, place l'ANCT dans une position d'acteur principal. La confiance dans l'agence et dans son bon fonctionnement est donc essentielle. Monsieur le secrétaire d'État, les préfets sont considérés comme les délégués territoriaux de l'ANCT ; comment comptez-vous corriger les petits problèmes pratiques constatés sur le terrain ? Cela pourrait-il passer par un renforcement du rôle et des pouvoirs dévolus

dont je vous donne quelques exemples : opération de revitalisation du territoire de Saint-Gaudens, à propos de laquelle je vous indique- je pense que vous le savez -que la candidature montée conjointement avec la commune, la communauté de communes et la DDT est lauréate d'un appel à projets

La création de cette agence apparaît d'autant plus justifiée aujourd'hui, à l'instant critique où notre pays se trouve et au regard des défis gigantesques qu'il aura à relever dans l'avenir. Dans la période d'épidémie que nous traversons, les collectivités sont aux avant-postes, dans des conditions d'autant plus difficiles que cette crise sanitaire est doublée d'une grave crise économique. La mise en oeuvre des mesures de distanciation sociale dans les lieux publics et les mairies et les achats supplémentaires de matériel rendus nécessaires par la crise ont eu un coût important, en particulier pour les petites communes. En outre, des investissements futurs sont à prévoir dans ce domaine. Je pense, par exemple, aux dispositifs de détection de virus dans les eaux usées des stations d'épuration gérées par les collectivités ; ceux-ci sont en train de faire leurs preuves à l'étranger et viennent de recevoir l'agrément qui autorise leur commercialisation en France. Il est évident que, après la fin de la pandémie de covid-19, la politique de prévention et de lutte contre les épidémies sera renforcée et remaniée, tant à l'échelon national qu'à Les collectivités seront nombreuses à vouloir agir dans ce domaine, pour protéger leur population. Mon propos n'est pas de faire peser toute la charge qui en résultera sur l'État, et encore moins sur l'ANCT,

C'est pourquoi je souhaiterais savoir si l'ANCT prévoit de mettre en place, à l'avenir, un dispositif spécifique d'aide aux collectivités dans le domaine de la lutte contre le risque épidémique.

va mettre en place un dispositif d'aide aux collectivités dans le domaine de la lutte contre le risque épidémique. C'est l'occasion pour moi de rappeler que, en tant qu'autorité de coordination interfonds,

tous ses travaux en collaboration avec Régions de France, avec les autorités de gestion des fonds européens et avec les services de l'État qui étaient directement concernés par ces fonds. Un dialogue en temps réel avec les services de la Commission a permis de bien faire remonter les problématiques et permet aujourd'hui de financer un certain nombre d'opérations.

Travailler, accéder à ses droits, engager des démarches administratives, étudier, se soigner devient pour beaucoup un défi insurmontable. Malgré les actions en faveur de l'inclusion numérique menées depuis une dizaine d'années, d'années, près de 13 millions de Français et de Françaises en demeurent exclus ; mais ce chiffre est, dit-on, largement sous-estimé. Ce qu'il faut bien appeler un échec est lié à l'absence de rationalisation de l'action publique. Le foisonnement de l'offre de médiation, avec des initiatives diverses, des situations différentes, des ressources dispersées et plusieurs niveaux de décisions, rend ces actions difficilement identifiables. preuve en est la faible utilisation du pass numérique. Éclatées, ces actions manquent de cohérence, d'organisation, de lisibilité et donc d'efficacité. La relance de notre pays ne peut faire l'impasse sur une véritable appropriation du numérique et de ses usages

de la transformation numérique et surtout de l'inclusion numérique. Concrètement, c'est d'un chef d'orchestre que nous avons besoin. L'ANCT pourrait jouer ce rôle, car ce sont les territoires qui permettront de mettre en oeuvre L'agence est-elle prête à assurer ce leadership pour, enfin, nous doter d'une stratégie cohérente, équilibrée territorialement et ciblée en direction des populations qui en ont besoin ? Si oui, comment ? La

des usages du numérique, est un élément extrêmement important dans la crise que nous traversons. L'action de l'ANCT porte sur le développement des infrastructures numériques dans les territoires, notamment ruraux, mais aussi sur la montée en compétences numérique des Français, ce

Pour autant, ce dont ont besoin les élus de la ruralité, c'est que ce type d'agence soit au rendez-vous en matière d'agilité et de réactivité, notamment dans leur capacité à mobiliser au plus vite les fonds du plan de relance.

de ne pas être entendus sur des sujets qui ont pourtant une résonance forte sur le terrain. Je pense, notamment, au développement de la téléphonie ou à certains axes de mobilité interdépartementaux, pour ne citer que les exemples auxquels je suis confronté dans mon département de l'Ardèche.

Hier, lors de l'audition de Mme la ministre de l'écologie, il a souvent été fait référence au Cerema comme point d'appui pour développer ces politiques. Je m'en félicite. Toutefois, le Cerema connaît une diminution continue de ses moyens humains et financiers, ce qui conduit à une fragilisation de ses compétences et obère ses capacités d'investissement. Les élus locaux ont rappelé à de nombreuses reprises la nécessité du Cerema comme outil d'ingénierie et d'expertise. Cette situation conduit à une contradiction entre les discours du Gouvernement sur la cohésion territoriale et la continuité d'un plan d'austérité, qui fragilise une expertise publique et indépendante au profit des territoires. En deux ans, le Cerema aura perdu 188 postes. Au-delà des chiffres, il faut considérer ce que les agents peuvent vivre et exprimer. L'analyse de la démarche « Cerem'Avenir » fait office de révélateur de l'ensemble des facteurs de risques professionnels auxquels sont exposés les agents : perte du sens du travail, surcharge de travail amplifiée, dégradation de la performance opérationnelle,

La convention signée entre l'État, l'agence et le Cerema ne prévoit aucune participation claire de l'ANCT au financement du Cerema. Enfin, comment comptez-vous garantir les moyens humains et financiers de ce centre tellement indispensable pour le développement de nos politiques publiques et pour le plein exercice de ces compétences ?

échanges entre l'ANCT et le Cerema sont réguliers, car ces établissements doivent se coordonner sur de nombreux sujets d'interaction. Vous savez quelles sont les capacités d'intervention du Cerema en ingénierie. C'est une condition aussi de la capacité de l'ANCT à agir au profit des collectivités qui nous sollicitent. Le Cerema est l'établissement de référence pour les questions territoriales, de gestion des risques-

des projets de territoire. Il existe des guides, des outils cartographiques de mise en valeur des données du territoire, des assistances territoriales, des assistances à maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre,

Cela dit, augmenter la charge des services tout en diminuant les effectifs, c'est un peu comme si, en mécanique, on augmentait les efforts sur un arbre en diminuant son diamètre ... Cela finit par casser.

même si elle avait été annoncée lors de la conférence des territoires ici même au Sénat, est la fille du grand débat qui a suivi la crise des gilets jaunes. Elle est aussi le syndrome français de la réponse à tout problème par une création nouvelle.

Pour être factuel, on peut enfin rappeler que l'ANCT est aujourd'hui encore une coquille assez largement vide, ou presque, sur nos territoires. Il est encore difficile de mobiliser des ressources de l'administration centrale et des opérateurs de l'État, trop éloignés, en complément de l'expertise des préfectures et des services déconcentrés de l'État, trop limitée. On ne peut pas réellement dire non plus que l'ingénierie locale est pleinement associée. L'ANCT est encore trop souvent une réponse verticale et centralisée au besoin d'ingénierie territoriale. Elle répond à une ambition légitime, mais sans réels moyens humains de la part de l'État. Elle offre à l'échelle départementale un espace de concertation et de partage utile, dont il faut renforcer l'efficacité. Elle n'associe pas assez les agences d'ingénierie départementales que les collectivités ont su mettre en place. en place. L'accompagnement des acteurs publics locaux, l'accélération de la vision territoriale, l'identification de réels choix structurels portés par l'agence sont pourtant des nécessités. Le diagnostic est juste, mais la réponse n'est ni suffisamment pragmatique, ni partagée. À l'heure du plan de relance au service des territoires ruraux, d'une relance qui mobilise tous les acteurs publics locaux, va-t-on enfin ajouter aux trois D annoncés le C de la confiance ? La confiance appelle à mettre au coeur de l'ANCT les élus locaux, pour territorialiser son action et la relance, ainsi que pour confirmer l'attractivité accrue de la ruralité. Le comité local de cohésion territoriale présidé par le préfet pourrait-il ainsi, monsieur le secrétaire d'État, être coprésidé par le président du conseil départemental ?

le secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Sautarel, vous m'interrogez sur le rôle que l'ANCT peut jouer dans la mise en oeuvre du plan de relance sur les territoires.

ont été interrogés par mes collègues sur les programmes de soutien aux communes, notamment ceux établis dans les territoires fragiles. Deux des propositions du rapport d'information de mes collègues Mme Josiane Costes et M. Charles Guené sur l'ingénierie territoriale et l'Agence nationale de la cohésion des territoires consistaient justement à favoriser l'émergence des projets lancés localement et à rendre prioritaire l'accompagnement dans les territoires les plus fragiles, vous avez rappelé à maintes reprises. Dans la continuité de leurs travaux, ma question porte sur le programme Petites villes de demain, à destination des communes qui comptent moins de 20 000 habitants et montrent des signes de fragilité, comme le rappelle la lettre d'engagement du programme. Entre 800 et 1 000 communes, partout en France, pourront être accompagnées dans le cadre de ce programme d'appui supervisé par l'agence. Monsieur le secrétaire d'État, le confinement de la population mis en place entre le 17 mars et le 11 mai 2020 s'est traduit par une contraction sans précédent de l'activité économique en France, ce qui a particulièrement touché le tissu économique de nos petites villes, composé en partie de commerces. Ainsi, les petites fragilités deviennent de plus en plus, hélas, de grandes vulnérabilités. Les élus locaux demeurent, comme toujours, en première ligne et se démènent chaque jour pour trouver des solutions. Ils attendent aujourd'hui un soutien de l'État, afin de redonner vie à nos petites bourgades. Ce sont trop souvent des communes oubliées, alors qu'elles contribuent au charme de notre pays. Les répercussions économiques des deux confinements seront-elles prises en compte dans la sélection des communes bénéficiaires de ce programme ? Sur quels critères sont identifiés les territoires vulnérables

M. Édouard Courtial. Monsieur le secrétaire d'État, la liberté d'habiter à la ville ou à la campagne est-elle encore une réalité dans notre pays ? La question se pose avec une acuité toujours plus accrue, tant les fractures territoriales se creusent. désertification médicale, administrative, scolaire et économique, les mobilités et l'accès au numérique sont parmi les défis que nos territoires ruraux doivent relever. Pour autant, ils ont de nombreux atouts, dont un cadre de vie qui convainc ou tente, surtout dans le contexte actuel, de nombreux citadins, non sans certaines difficultés d'adaptation. L'Agence nationale de la cohésion des territoires, dont le titre même est une promesse, doit donc être à la pointe de ce combat, qui engage notre avenir. Un an après le vote de la loi, dresser son bilan serait prématuré et les réserves qui ont présidé à sa création restent d'actualité, même si le Gouvernement, auditionné au Sénat il y a quelques jours, a voulu apporter des garanties. de créer un outil permettant de travailler en tandem avec les territoires pour les accompagner, pour les aider à développer leurs projets et pour coordonner l'action de l'État avec celle des collectivités territoriales, il serait inutile et

L'ANCT doit donc d'abord être réellement au service des territoires et s'appuyer avant tout sur le bon sens des élus locaux, qui sont au contact des réalités du terrain. Elle doit ensuite ne pas nuire aux collectivités en accaparant des ressources qui leur seraient destinées et fortement utiles, y compris pour faire face à l'épidémie que nous traversons. enfin ne pas se substituer aux collectivités territoriales, qui, en la matière, oeuvrent sans relâche et avec détermination ; je pense, notamment au conseil départemental de l'Oise. Faute de prendre en compte ces avertissements, l'ANCT créerait des espoirs déçus, qui alimenteraient encore davantage la défiance d'élus locaux se sentant de plus en plus dépossédés, aussi bien en termes de compétences que de moyens, alors que les attentes de leurs administrés n'ont jamais été aussi importantes. Le premier vrai test est donc devant nous.

Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur la prise en compte des élus locaux dans l'ensemble des politiques relatives à l'ANCT.

vingt-cinq propositions. Nous avons souhaité mettre en parallèle les ambitions de l'ANCT et la réalité des besoins de nos territoires en matière d'ingénierie, dans leur diversité. Nous avons pu, à cet égard, rappeler la volonté originelle du législateur et, par là même, ébaucher un débat fructueux avec l'administration, qui mettait en oeuvre cette nouvelle structure. Nous étions et nous sommes assez confiants sur la mission principale de l'ANCT, qui a proposé de réorganiser l'action de l'État et la conduite de sa politique territoriale. Toutefois, nous avons insisté

Cette inclination nécessite la réalisation d'un état des lieux et la mise en oeuvre de gouvernances locales autour du préfet. Malgré les difficultés liées à la pandémie que nous comprenons bien, où en êtes-vous dans cette démarche, tant sur le plan structurel que par rapport au plan de relance ? ? Enfin, lors de l'examen des crédits de l'outre-mer, notamment au regard du logement, nous avons constaté une grave sous-consommation des crédits de paiement alloués, et cela, nous ont dit nos collègues, en raison du manque d'ingénierie.

Cette période de flottement, que j'espère aussi courte que possible, peut expliquer l'incompréhension et la perplexité des élus face aux missions de l'Agence. En effet, à ce stade, le rôle opérationnel de l'Agence tant dans la conception

tardivement. Les crédits de l'enveloppe de l'ANCT dédiée à l'ingénierie territoriale, d'ailleurs sous-consommés en 2020, devraient être affectés exclusivement aux projets lancés par les collectivités, notamment par les plus fragiles, tout en assurant un équilibre entre les villes et les territoires ruraux. La transparence sur ces données serait la bienvenue. Le circuit de la décision doit être clarifié et cette lourde tâche revient au pouvoir réglementaire.

permettant au nouvel organisme de répondre aux attentes des collectivités territoriales et d'assurer pleinement sa mission de coordination des actions et des projets des autres services et opérateurs de l'État. Il conviendra également qu'il soit doté, tant au plan national que local, des ressources suffisantes. » Les critiques relatives à la lisibilité de la coordination entre les différents opérateurs doivent être prises en compte.

départementales des territoires. Nous pourrions ainsi gagner en efficacité dans l'instruction des dossiers. Pour conclure, je tiens à remercier, au nom du groupe du RDSE, l'ensemble des collègues de leur participation à ce débat et de la qualité de leurs interventions.

de faire de l'Agence nationale de la cohésion des territoires le bras armé de la lutte contre la fracture territoriale ; tel était l'esprit initial de la proposition de loi que nous avions portée. Nous en avons terminé avec le

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

De quoi nous réjouir, certes, mais, comme le dit l'adage, il y a loin de la coupe aux lèvres et la réussite de notre conversion à l'hydrogène nécessite non seulement une ambition, mais également des préalables et des conditions de réussite. L'ambition, c'est celle de développer une filière vertueuse, capable de placer notre pays en tête de la course qui s'est engagée pour la conquête du leadership dans le développement de l'hydrogène, face aux deux géants concurrents : la Chine et les États-Unis. une filière, cela signifie créer les conditions pour que s'exprime la demande. Or, on le sait, pour le moment, le recours à l'hydrogène comme source d'énergie coûte cher. Il faut donc agir à grande échelle et impulser une massification de la demande, au travers des secteurs les plus consommateurs d'énergie : la mobilité et l'industrie. La conscience de la nécessité d'une transition énergétique est aujourd'hui largement partagée, mais il faut convaincre et, pour cela, il faut accompagner et garantir. J'y reviendrai.

des préalables incontournables. Tout d'abord, si la France veut être leader, elle ne peut y arriver seule, cela n'aurait aucun sens.

C'est précisément là que se niche l'une des premières conditions de notre succès. Pour réussir, le projet français doit s'inscrire pleinement dans cette stratégie européenne. Or des inquiétudes se font déjà Notre hydrogène « bas carbone » sera majoritairement « nucléarisé », ce qui ne plaît pas à certains de nos partenaires européens, comme l'Allemagne, qui fait le choix d'un hydrogène strictement renouvelable, importé massivement de pays où la production de renouvelable est abondante et peu chère. La Commission semble privilégier une approche similaire. Il faudra donc veiller à ce que la France ne soit pas exclue des outils de politique publique ni des financements Cette divergence est d'autant plus préoccupante que la Commission semble vouloir imposer l'éligibilité de la production d'hydrogène à la taxonomie verte, un seuil d'émissions de gaz à effets de serre difficilement atteignable pour les producteurs français, en particulier ceux qui recourent au solaire ou à l'électricité.

il serait illusoire, et même dangereux, de vouloir développer le recours à l'hydrogène dans tous les secteurs. La France fait le choix d'axer la conversion à l'hydrogène pour décarboner deux secteurs essentiels : l'industrie et la mobilité. Les applications à l'échelle des particuliers sont possibles, mais, d'une part, les coûts demeurent prohibitifs et, d'autre part, les évolutions technologiques permettant de les envisager en sont encore, pour la plupart, au stade expérimental. il ne faudrait pas qu'un secteur vienne en concurrencer un autre, après les nombreux efforts déjà consentis, par exemple par les constructeurs automobiles, pour dynamiser la voiture électrique ou hybride. Là encore, les conditions de la réussite doivent être créées. Ainsi, les efforts des industriels doivent être encouragés et récompensés. On le sait bien, tout changement d'importance doit être accompagné de mesures incitatives. En ce qui concerne les transports, notre pays fait le choix de concentrer son action sur les véhicules lourds et sur la transformation du transport de passagers et de marchandises. Pour les poids lourds, une prime à la conversion et une prime à l'acquisition seront mobilisées. Le secteur ferroviaire se mobilise également, quatre régions s'étant engagées dans l'achat de trains express régionaux (TER) circulant à l'hydrogène. Viendront ensuite les navires et l'aéronautique, l'objectif étant de produire un avion neutre en carbone en 2025. d'une feuille de route dense, avec des objectifs d'envergure qui ne seront atteignables que si notre pays investit et s'investit dans le champ de l'innovation et dans la recherche et développement. l'objet, d'une part, de l'appel à projets Briques technologiques et démonstrateurs, doté, jusqu'en 2023, de 350 millions d'euros pour l'amélioration des composants et systèmes liés à la production et au transport de l'hydrogène du programme prioritaire de recherche sur les applications de l'hydrogène, engageant 65 millions d'euros pour préparer la future génération des technologies de l'hydrogène, qu'il s'agisse des piles, du stockage ou encore des électrolyseurs. En complément nécessaire au bouclage de cette filière vertueuse, un budget de 30 millions d'euros a été affecté à la création, en 2021, de campus des métiers et des qualifications pour drainer la formation et l'enseignement supérieur, afin que notre pays se dote des professionnels qualifiés capables de faire vivre cette industrie nouvelle. sur le papier, tout est réuni pour que cette initiative soit un succès, mais, bien évidemment, des points de vigilance existent et ils sont loin d'être négligeables. J'ai évoqué l'un des principaux, l'articulation de notre stratégie avec celle de l'Europe.

vigilants également sur le risque de bulle financière. Des milliards d'euros sont sur la table et ils aiguisent les appétits ; et grands groupes se précipitent pour collecter les financements publics. Attention donc à la spéculation et aux opportunistes, qui vendent leur projet avant même d'avoir produit quoi que ce soit

vert. Certains pays seront alors tentés de compléter le dispositif européen en construisant des dispositifs, dans des pays où l'énergie renouvelable est abondante et peu chère, comme en Ukraine ou dans les pays d'Afrique du Nord, et en rapatriant ensuite

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, l'hydrogène est l'une des grandes révolutions technologiques de ce début de siècle ; il représente une opportunité stratégique pour contribuer à la décarbonation de notre économie, particulièrement dans l'industrie et la mobilité lourde.

Notre pays a fait très tôt le pari du soutien à cette filière d'avenir : en 2018, Nicolas Hulot annonçait un premier plan Hydrogène, doté de plus de 100 millions d'euros, mobilisés le programme d'investissements d'avenir

Une France neutre en carbone, ce sera d'abord une France qui améliore la santé de ses habitants. La crise sanitaire que nous vivons le rappelle

construire des usines d'électrolyseurs et de composants clés dans nos territoires, de faire émerger et de déployer sur l'ensemble du territoire des solutions d'hydrogène décarboné. Nous visons

Cet investissement massif sera gage de notre succès, vous l'avez dit ; il faut absolument aller vite et fort, pour déployer les marchés les plus matures, soutenir la recherche et l'innovation sur les segments d'avenir, en pensant notamment aux nouveaux usages industriels et au stockage d'énergie.

l'État a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour aider à l'émergence de la mobilité à l'hydrogène dans le ferroviaire, pour lever tous les verrous techniques et organisationnels et pour préparer la mise en service des premières rames d'ici à cinq ans. ans. Quatre régions pionnières de l'hydrogène et du TER de demain ont été retenues : le Grand Est- en tant que Haut-Marnaise, je m'en félicite -, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, suivie d'une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

à discuter, avec plusieurs partenaires, de la place de l'hydrogène dans la décarbonation des réseaux énergétiques et du retour d'expérience sur la gestion des réseaux par injection d'hydrogène pour décarboner les énergies

À l'issue de ces six années d'expérimentation, les onze partenaires sont unanimes : la mise en oeuvre du projet Grhyd, véritable test sur le terrain, a permis de démontrer la pertinence technique de l'utilisation d'une énergie fondée sur l'hydrogène vert pour les habitations. En bref, ce projet a permis de valider les technologies et l'efficacité du, en toute sécurité, et d'évaluer les bénéfices environnementaux d'une telle filière. Tous ces éléments seront de précieux enseignements pour la suite, lors du développement du à l'échelle locale et nationale, voire internationale. Quelque 100 logements et la chaufferie d'un centre de soins ont été alimentés par un nouveau gaz, composé d'une part variable d'hydrogène- à hauteur de 20 % au maximum -et de gaz naturel, avec des résultats plus que pertinents en termes de réduction des émissions de polluants atmosphériques. Ce projet est un succès, même s'il reste quelques champs à examiner avant de pouvoir généraliser l'injection d'hydrogène dans le réseau de gaz naturel. La question de l'acceptabilité sociale de l'hydrogène est l'une des clés de la réussite du déploiement de ce gaz dans nos maisons et dans notre vie quotidienne. La participation citoyenne aux discussions sur l'hydrogène et la diffusion des connaissances scientifiques auprès du public constituent donc des enjeux essentiels. À cet égard, l'expérience menée avec les habitants du petit village de Cappelle-la-Grande est riche d'enseignements.

Comme pour de nombreux projets, la conception en amont, ainsi que les procédures réglementaires d'autorisation devront être particulièrement soignées. Elles devront favoriser la mise en relation des acteurs, dont les futurs consommateurs d'hydrogène, pour que se mette en place un véritable projet de territoire ; elles devront aussi prendre en compte les enjeux environnementaux, typiquement la consommation d'eau des électrolyseurs, et veiller à une concertation de qualité avec les riverains et les collectivités locales. Le projet Grhyd que vous évoquez a été soutenu par l'Ademe. Il vise à réaliser un premier démonstrateur d'injection d'hydrogène dans le réseau de gaz naturel et à développer l'acceptabilité locale. Une aide de près de 5 millions d'euros sur 15 millions d'investissements a ainsi été apportée à cet effet. Comme vous le soulignez, c'est une première étape pour l'injection ; de nombreux autres projets de

Pour cette transition énergétique, elle mise sur un volet hydrogène très ambitieux. Pionnière, elle est labellisée Territoire d'hydrogène depuis 2016. Son plan de développement Hydrogène vert destiné à favoriser de nouvelles productions et de nouveaux usages est doté de 150 millions d'euros d'ici à 2030 et pourrait générer jusqu'à un milliard d'euros d'investissements. Déjà, les projets HyDéO, HyPort à l'aéroport de Toulouse-Blagnac ou encore Hyd'Occ à Port-La-Nouvelle sont lancés. L'achat de trois trains hybrides à hydrogène est programmé, ce qui est une grande première. La région prévoit aussi la mise en circulation de 3 250 véhicules à hydrogène d'ici à 2030. dans l'Hérault, une station de distribution va s'installer. À Béziers, grâce aux électrolyseurs développés par le Commissariat à l'énergie atomique, un site produira en 2021 de l'hydrogène vert trois à quatre fois moins cher qu'aujourd'hui. Dans ces conditions, cette énergie devient très compétitive face aux hydrocarbures et aussi en termes de bilan carbone. Notre collègue Éric Gold compte dans son département un champion industriel, Michelin, qui est engagé dans la filière hydrogène et qui entend devenir l'un des leaders mondiaux de la mobilité. Ce n'est sans doute pas un hasard si la région Auvergne-Rhône-Alpes concentre 80 % des acteurs de la filière hydrogène en France. Pour relever ce défi, il faudra cependant résoudre une équation qui reste encore floue, celle de l'équipement de notre territoire en stations de distribution pour approvisionner les véhicules grand public en hydrogène.

et les opérations locales de déploiement cofinancées par l'État et les collectivités territoriales. D'ailleurs, l'appel à projets Briques technologiques permettra, entre autres, de soutenir les porteurs de projets pour industrialiser la production de stations de ravitaillement. L'appel à projets Écosystèmes territoriaux permettra quant à lui de soutenir notamment les infrastructures de distribution d'hydrogène à l'intention des flottes professionnelles. À plus long terme, d'ici à une dizaine d'années, quand les procédés de production des différents systèmes seront devenus très compétitifs, l'hydrogène pourra éventuellement s'adresser aux véhicules destinés à l'usage des particuliers.

qui nous donne l'occasion d'insister sur l'importance du développement et du maintien de l'industrie sur notre territoire. Si l'hydrogène comme solution de remplacement et comme moyen de réduire l'empreinte carbone des carburants est prometteur, il pose encore un certain nombre de questions.

l'automobile et le train. Aussi, pour que la France devienne un champion de l'hydrogène, des investissements massifs doivent être réalisés. Surtout, une filière industrielle complète et publique doit impérativement être constituée, tant en termes de recherche et de développement que de production et de réalisation d'installations. La constitution d'une filière publique est nécessaire pour éviter un gaspillage de l'argent public. C'est d'autant plus le cas que, à l'heure actuelle, la production d'hydrogène est majoritairement réalisée à partir de gaz naturel, une tonne d'hydrogène étant produite pour dix tonnes de CO2 émis.

d'ici à 2022 dans le plan de relance, quelle stratégie industrielle intégrée comptez-vous mettre en place pour que naisse une véritable filière stratégique et de services permettant de produire de l'hydrogène de manière propre ? Sur quel opérateur allez-vous vous appuyer pour la construire ? La parole est

pour développer et déployer des solutions de mobilité lourde sans émission. Les 7 milliards d'euros de soutien public d'ici à 2030 vont permettre d'alimenter une stratégie d'offre et de demande équilibrée.

D'autre part, et en parallèle, la stratégie nationale a pour ambition de soutenir le déploiement sur le territoire d'infrastructures de production et de distribution d'hydrogène pour décarboner l'industrie et la mobilité lourde.

de certains segments de mobilité, comme les camions. Enfin, un appel à projets Briques technologiques et démonstrateurs, destiné à soutenir l'innovation, a été lancé le 14 octobre. Financé à hauteur de 350 millions d'euros, il vise à développer et à améliorer les composants et les systèmes liés à la production et au transport de

Dans ce contexte, l'un des enjeux environnementaux des dix prochaines années est de décarboner l'industrie et la mobilité lourde. de ce point de vue, l'hydrogène dispose de nombreux atouts, même si ses débuts sont encore timides, faute d'une industrialisation à grande échelle. Toutefois, une approche durable de cette énergie implique de remplacer l'hydrogène dit « gris »- sa production dépend d'énergies fossiles et génère des émissions de gaz à effet de serre -par de l'hydrogène décarboné.

ou l'hydroélectricité. D'ores et déjà, des collectivités ont franchi le pas ; c'est le cas de la communauté d'agglomération paloise qui a, par exemple, mis récemment en service une flotte de bus équipés d'une motorisation à hydrogène, dont la production est issue de l'hydroélectricité certifiée d'origine, provenant des barrages de la Société hydroélectrique du Midi situés dans la vallée pyrénéenne voisine. Le choix de l'hydroélectricité, qui n'est pas une énergie renouvelable intermittente, contrairement au photovoltaïque et à l'éolien, est tout à fait pertinent pour verdir la production d'hydrogène. Malheureusement, l'hydroélectricité est rare

comme au développement économique des territoires. Pour ces raisons, la petite hydroélectricité fait l'objet, au même titre que plusieurs autres filières d'énergie renouvelable, d'un soutien clair du Gouvernement à la fois un arrêté tarifaire et des appels d'offres périodiques lancés par le ministère de la transition écologique. Toutefois, la multiplication de ces de ces installations dans les cours d'eau peut avoir, par effet de cumul, des effets importants sur l'environnement. En effet, les seuils fragmentent les cours d'eau et empêchent, plus ou moins fortement, le déplacement des espèces qui est nécessaire à l'accomplissement de leur cycle de vie. Ils peuvent également ralentir les eaux qui se réchauffent alors plus vite l'été, perdent en oxygène et créent des habitats de milieux stagnants, lesquels favorisent malheureusement des espèces moins exigeantes et moins diversifiées, parfois incompatibles avec le bon état des cours d'eau. Ces retenues peuvent en outre ennoyer des habitats, qu'il faut ensuite reconquérir pour restaurer une biodiversité aquatique. Le développement de la petite hydroélectricité devra donc être sélectif et limité et faire l'objet d'une réflexion à l'échelle du cours d'eau sur la proportionnalité des impacts par rapport à la production électrique générée. souligne aussi que, compte tenu de la taille et de la puissance de ces installations, elles ne pourront jouer qu'un rôle limité dans l'atteinte des objectifs nationaux. La production d'hydrogène nécessitant des puissances relativement importantes, le couplage

est dans le mix électrique. À cet égard, l'hydrogène vert est un vecteur de premier plan pour réussir la transition énergétique. L'hydrogène peut être produit par électrolyse de l'eau, grâce à l'électricité produite en période creuse en provenance d'installations d'énergies renouvelables- éolien, photovoltaïque ... C'est alors de l'hydrogène de l'hydrogène vert, par essence renouvelable et décarboné, mais aussi facilement stockable puisque c'est un gaz. Si les propositions législatives de l'Union européenne pour une Europe climatiquement neutre sont en cours, plusieurs pays membres ont déjà demandé à la Commission de garantir la traçabilité de l'hydrogène renouvelable. Pour être en accord avec nos engagements climatiques pris dans le cadre de l'accord de Paris, nous devons produire de l'hydrogène vert. Développer une filière compétitive en France est donc non seulement une nécessité écologique, mais aussi une question de souveraineté. Pour être compétitive en la matière, la France doit avoir un plan ambitieux et cohérent de structuration de cette filière. C'est un défi en raison du coût élevé de la production par électrolyse de l'eau et de la chute du prix des énergies fossiles, deux éléments qui favorisent la production d'hydrogène par vaporeformage. Nous devons être en mesure de rendre le prix de l'hydrogène vert suffisamment attractif pour favoriser les investissements dans les infrastructures. Nos territoires sont la clé du dynamisme et de l'équilibre de cette filière, dont le potentiel est non négligeable pour le marché de l'emploi. C'est depuis les territoires, avec les collectivités, que devront se développer les projets qu'il faut dès lors accompagner par une stratégie nationale simplifiée et une politique forte C'est ainsi que nous entrerons dans une dynamique vertueuse, condition de l'équilibre financier de la filière. Ma question porte sur les électrolyseurs. Où en est-on dans le développement de cette technologie d'avenir ? Des fabricants français sont-ils d'ores et déjà prêts à se lancer dans l'aventure ?

l'électrolyse sera privilégiée, l'objectif étant d'atteindre une puissance installée de 6,5 gigawatts sur le territoire national d'ici à 2030. L'un des objectifs de la stratégie est de positionner notre pays, à travers ses industriels, comme un leader mondial dans la production d'électrolyseurs performants de bon rendement, à des coûts permettant de les diffuser largement sur les marchés de la filière hydrogène. Clairement, la stratégie nationale a vocation à favoriser l'implantation sur le territoire national de d'électrolyseurs. L'appel à projets Briques technologiques et démonstrateurs a ainsi vocation, entre autres, à soutenir les industriels dans leur effort d'industrialisation d'électrolyseurs, du prototype

Il présente l'avantage d'autoriser les pouvoirs publics à soutenir les participants au-delà du stade de la recherche, en finançant le passage des innovations à la production. Il doit contribuer de manière concrète, claire et identifiable à un ou plusieurs objectifs de l'Union

; déploiement de flottes de véhicules lourds utilisant notamment l'hydrogène- bus, autocars, camions et véhicules de collecte des déchets - ; soutien à des projets visant à améliorer la production de composants stratégiques afin d'alimenter la chaîne d'approvisionnement des futurs véhicules en grande série ; soutien aux efforts de recherche pour les différents modes de transport-

Je vous remercie

Madame la secrétaire d'État, les enjeux de la relance nous obligent à imaginer un avenir différent. Les plans français et européens proposent une croissance verte et l'hydrogène, dans lequel je crois depuis longtemps, y tiendra une place principale.

Chacun doit prendre sa part. L'argent public ne sera efficace que si l'argent privé est aussi investi dans des projets d'avenir, qui sont par ailleurs coûteux. Les effets de levier seraient vertueux et cela donnerait du souffle à l'État, dont l'endettement explose.

d'un moyen d'investir son épargne, des plateformes numériques, dans des entreprises françaises, en particulier dans notre tissu de PME-TPE. Cela peut prendre la forme de financements interentreprises ou concerner des investisseurs particuliers ou des personnes morales. Madame la secrétaire d'État, envisagez-vous de garantir et d'accompagner l'intégration de telles plateformes de financement participatif dans la stratégie hydrogène de la France ?

des acteurs importants aux côtés des collectivités et des financeurs régionaux, qui sont également très investis dans la croissance verte. Beaucoup reste à faire, mais je suis très confiante dans l'avenir de ces projets de territoire localisés, qui font sens et permettent

L'hydrogène est une énergie de stock et non une énergie de flux, comme l'électricité. C'est là tout son intérêt : elle peut être associée à des énergies intermittentes, comme le solaire et l'éolien. Avec cette stratégie, nous avons une chance importante de faire de l'hydrogène un vecteur de la transition énergétique. Cependant, soyons vigilants et précis afin d'éviter les écueils de maintes politiques présentées comme étant très vertes. Aujourd'hui, plus de 95 % de l'hydrogène produit est un hydrogène gris, c'est-à-dire produit à partir d'énergies fossiles. L'intérêt écologique de cet hydrogène pour les mobilités est donc nul, pour ne pas dire négatif. Il ne faut donc pas développer la consommation d'hydrogène sans nous être au préalable assurés qu'il pourra être produit à partir d'énergies renouvelables. La technique de production par électrolyse est une technologie tout à fait intéressante, dès lors qu'on utilise des énergies renouvelables. Qu'en est-il du bilan écologique du dans son ensemble ? Je pense en particulier aux électrolytes et aux piles à combustible.

du comité de pilotage chargé de l'élaboration du plan de programmation des ressources minérales de la transition bas carbone. Les technologies d'électrolyseurs ont aujourd'hui recours à des matériaux dont la criticité est jugée faible à modérée par le Bureau

de protons. Plus largement, la Commission européenne a prévu de lancer une action de surveillance pour s'assurer du bon approvisionnement des matériaux nécessaires à la production des éléments de la chaîne de valeur des technologies de l'hydrogène.

La filière de l'hydrogène est séduisante, et il faut pousser la recherche, bien entendu, mais ne mettons pas, une fois encore, tous nos oeufs dans le même panier. N'oublions pas que la sobriété et l'efficacité énergétiques sont à la base de la transition écologique. La parole est à Mme Catherine Fournier.

Compte tenu de son mix électrique faiblement émetteur de CO2, la France dispose d'atouts pour produire cet hydrogène décarboné. Je vous alerte cependant sur la matière première de fabrication, à savoir l'eau, qui est une ressource essentielle. Sa gestion industrielle devra être adaptée. Il reste l'hydrogène bleu, fabriqué à partir de la technique de pyrolyse de gaz naturel, gaz essentiellement composé de méthane. Il représente une ouverture pour la gestion des déchets de l'agriculture et des centres de traitement. L'hydrogène est un volet du plan de relance. Il s'agit de positionner la France comme championne de sa fabrication, mais ne nous voilons pas la face : devenir leader, c'est développer une stratégie agressive en matière d'innovation,

en particulier par électrolyse, et à la baisse des coûts par effet d'échelle, grâce à des électrolyseurs moins chers et à des usines d'électrolyse plus importantes, nous comptons bien réduire cet écart le plus fortement possible. égard, des perspectives de réduction bien en deçà du facteur 3 ou 4 que vous évoquez nous semblent crédibles d'ici à quelques années. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ni même du Gouvernement. C'est le point de vue d'experts et d'industriels très impliqués dans le développement de ces filières. votre question, il faut en effet concilier réussite de la décarbonation de nos économies, nationale et européenne, et maintien de la compétitivité, en particulier dans les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale. Dans le cadre des discussions actuelles sur le renforcement de l'objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030, nous avons proposé de travailler opérationnellement à la mise en place d'un mécanisme dit d'ajustement carbone

considèrent aujourd'hui cette proposition très favorablement. Nous devrions entamer en 2021, sous l'égide de la Commission européenne, l'écriture d'un texte législatif opérationnel sur une refonte du dispositif, dit ETS, de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ce qui nous offre des perspectives assez rassurantes.

une forte impulsion aux transports, et singulièrement à la filière hydrogène. Le tourisme fera partie des secteurs clés de la relance de l'économie mondiale. Comme il apparaît illusoire de vouloir cesser tout déplacement aérien dans un monde globalisé, il est indispensable de verdir les déplacements en utilisant une énergie moins polluante, comme l'hydrogène. L'Allemagne a très vite mesuré cette urgence. Pour relancer ce secteur, elle a décidé de consacrer 9 milliards d'euros aux transports et à la filière hydrogène.

Certaines régions anticipent déjà ces changements. La région Occitanie a ainsi été pionnière en matière de commandes de matériel roulant à hydrogène auprès d'Alstom pour équiper ses TER. Elle est aujourd'hui rejointe par d'autres régions.

permettre à la France d'être à la pointe de la production d'hydrogène renouvelable. Néanmoins, comment vont se décliner concrètement les 7 milliards d'euros du plan hydrogène ? Quels secteurs vont en bénéficier en priorité ? Pouvez-vous nous présenter l'échéancier précis de ces investissements ?

l'hydrogène constitue une piste stratégique, vous l'avez dit, pour réussir la transition vers une économie zéro carbone, en particulier dans le secteur de l'industrie et de la mobilité lourde. En se dotant d'une stratégie hydrogène ambitieuse pour accélérer le déploiement des filières de production et d'utilisation de l'hydrogène par électrolyse,

Nous avons également beaucoup avancé sur la définition d'un mécanisme de soutien à la production d'hydrogène décarboné et même commencé les discussions avec la Commission européenne pour sa notification comme aide

325 millions d'euros

Une énergie sans émission de CO2 est intéressante, à l'heure où la question de l'enfouissement du gaz carbonique fait débat. Les régions ont saisi ces capacités de décarbonation pour l'industrie et les mobilités. Elles ont été pionnières dans le soutien à l'hydrogène et portent des projets de déploiement de solutions adaptées. la région des Pays de la Loire, sous l'impulsion de sa présidente, Christelle Morançais, débloquera 100 millions d'euros d'ici à 2030 pour développer l'hydrogène et en faire une filière d'excellence. Dans les mobilités, la logistique, des projets émergent et gagnent en maturité, témoignant d'une ambition industrielle de long terme.

Le Gouvernement avait par exemple dilué sur trois ans les engagements du plan hydrogène de Nicolas Hulot, juste après la démission de ce dernier. Nombreuses sont les filières industrielles que l'État a souhaité développer pour la transition énergétique, sans que cela aboutisse. les régions s'engagent, l'État doit lui aussi le faire à long terme. Le développement de l'hydrogène doit s'inscrire dans une vision d'ensemble de l'évolution du système énergétique et des usages associés.

à la demande en consommation. En 2020, certes du fait de la crise, la chute du marché de gros de l'énergie a conduit à plusieurs reprises à des prix négatifs. Ce phénomène risque de se reproduire en raison de la part croissante du renouvelable non pilotable dans le mix énergétique. Le stockage de l'électricité par le biais de l'hydrogène est un levier qu'il devient donc urgent d'activer, mais les performances et les capacités ne sont pas encore au rendez-vous. Dans sa récente fiche technique, l'Ademe relève que le rendement de la chaîne de l'hydrogène est à l'heure actuelle de 23 % entre l'électricité induite dans l'électrolyseur et celle qui est restituée par la pile à combustible, alors qu'il est de 70 % pour les batteries. Sans opposer les deux modes de stockage, cette note montre le chemin qu'il reste à parcourir. Pour relever ce défi, non seulement des moyens financiers, mais aussi une organisation qui évite la dispersion et le saupoudrage des crédits, souvent ventilés entre de multiples équipes à la suite des appels à projets.

Houllegatte, l'échelon européen est crucial pour le développement de la filière de l'hydrogène. À cet égard, la publication de la stratégie européenne en juillet 2020 est une première étape très positive. Celle-ci identifie la filière électrolyse comme une filière d'avenir et porte un objectif ambitieux de 40 gigawatts en 2030. L'enjeu est de construire des champions européens

la stratégie nationale de la France rejoint sur de nombreux points les fondamentaux de la stratégie européenne. Les discussions sont actuellement en cours avec d'autres États membres pour mettre en place des projets importants d'intérêt européen commun, des des projets partenariaux en vue de soutenir les industriels français et européens de la filière de l'hydrogène afin de leur permettre d'investir plus massivement quand cela est nécessaire. Ces projets seront notifiés à la Commission européenne. La première réunion a eu lieu à haut niveau entre la Chancelière allemande et le Président de la République afin d'identifier les secteurs clés de cette coopération coopération : la production d'électrolyseurs, les composants clés et des projets de décarbonation, notamment. Ces grands axes se traduiront également par l'émergence de projets communs entre industriels. Ceux-ci seront suivis de près par les ministères de chaque pays pour faciliter leur déploiement, en particulier en combinant des soutiens financiers européens et nationaux. En complément, une feuille de route « recherche » a également été construite avec l'Allemagne sur l'énergie durable. Un appel à projets sur les énergies 2018, l'hydrogène étant identifié comme un secteur clé. Les dispositifs français viennent en complément des dispositifs européens, notamment l'Ademe. Cette articulation des différents dispositifs

de cohérence. La parole est à M. Stéphane Piednoir. Madame la secrétaire d'État, si nous voulons inscrire l'hydrogène dans notre futur mix énergétique, il nous faut trouver le moyen de le produire de la façon la plus vertueuse possible sur le plan environnemental.

mais la question de la source d'électricité utilisée se pose de manière cruciale, car elle conditionne la couleur environnementale de l'hydrogène. L'abandon des énergies fossiles ne peut se concevoir que si nous les remplaçons par des solutions faiblement émettrices de gaz à effet de serre. Certains pensent associer les énergies renouvelables aux électrolyseurs, mais cela ne pourra pas constituer un remède miracle, en raison de leur caractère intermittent, qui ne peut objectivement pas être occulté. Alors, faisant fi de quelques positions dogmatiques, nous devons être pragmatiques pour atteindre nos objectifs environnementaux, en nous appuyant sur des technologies totalement maîtrisées et faiblement émettrices de CO2. Ce débat est donc, me semble-t-il, une très bonne occasion de nous interroger sur la complémentarité entre le nucléaire et la production d'hydrogène décarboné. Je ne méconnais pas les griefs à l'encontre de l'atome, mais il devrait y avoir un consensus sur cet outil industriel, dont l'investissement est largement amorti. amorti. Par son caractère pilotable, il est un formidable atout pour équilibrer notre réseau électrique lors de fortes fluctuations de production des

jaune ? La parole est à Mme la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Piednoir, afin que l'hydrogène apporte son plein potentiel pour la décarbonation de l'économie, des usages nouveaux, comme la mobilité lourde ou la production de chaleur à haute température pour l'industrie,

La Commission européenne est convaincue qu'il est nécessaire de recourir à d'autres modes de production d'hydrogène bas carbone que la seule production d'hydrogène renouvelable, et ce principalement pour réduire rapidement les émissions des installations de production d'hydrogène existantes, et de soutenir l'adoption, en parallèle, et dans l'avenir, de l'hydrogène renouvelable. Avec des objectifs de production d'hydrogène décarboné à hauteur de 6,5 gigawatts et 600 000 tonnes à l'horizon 2030, la stratégie nationale de la France rejoint sur de nombreux points les fondamentaux de la stratégie européenne. En ce sens, la production d'hydrogène par électrolyse fera appel aux productions d'énergie renouvelable, comme à la production bas carbone qu'offre actuellement le mix électrique français. Nous avons, pour ce faire, des objectifs et une feuille de route, à la fois

Il semble que le Gouvernement voulait nous ménager un effet de surprise. À la bonne heure ! J'ai parfois tendance à penser que le covid-19 peut avoir du bon ... Une part très importante de cette enveloppe cible la décarbonation de l'industrie et la production d'hydrogène. Je m'en réjouis, mais pour bien développer l'économie de l'hydrogène et préserver notre souveraineté, il faut parvenir à faire émerger simultanément ses usages. Ce plan de relance doit aussi être l'occasion de les diversifier. Madame la secrétaire d'État, vous aurez compris que ma question porte sur les moyens et dispositifs mis en oeuvre par la France pour rester dans la course de la mobilité hydrogène.

Plusieurs projets sont portés aujourd'hui par de petites structures à l'échelle locale, mais c'est loin d'être suffisant pour générer une demande à la hauteur de l'offre qui existera dans quelques années. Si la demande n'émerge pas en France, l'offre sera bel et bien présente, mais elle viendra de l'étranger. Il faut soutenir l'émergence d'une filière industrielle française, sans reproduire les erreurs commises dans le passé pour les batteries ou les panneaux solaires. Des milliers d'emplois en dépendent, notamment dans le secteur automobile. Quelles initiatives, ou mesures, l'Europe et le Gouvernement prennent-ils pour stimuler cette filière, qui pourrait permettre la réindustrialisation des territoires oubliés ? Je pense notamment à de possibles souplesses administratives, qui rendraient le cadre réglementaire plus incitatif, mais aussi à des mécanismes de soutien public, ou encore à une taxation du carbone aux frontières européennes, à rendre plus compétitif l'hydrogène face aux hydrocarbures. Des discussions sont-elles engagées entre le Gouvernement et la Commission européenne ? En présentant le plan hydrogène, au début de septembre, Bruno Le Maire expliquait que le déclassement français, c'était le renoncement des élites.

le plus rapidement possible. Il s'agit, comme vous l'avez dit, de concilier la réussite de la décarbonation de notre industrie nationale et européenne avec le maintien de notre compétitivité dans les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale.

Madame la secrétaire d'État, filière d'avenir et alternative sérieuse aux énergies fossiles, l'hydrogène se situe à un moment stratégique de son développement, qui nécessite l'engagement de tous pour renforcer la dynamique. À cet égard, la place des territoires est essentielle. Il faut construire au plus vite un écosystème territorial performant pour ne pas risquer, comme nous l'avons malheureusement subi dans d'autres secteurs, la perte de notre indépendance, avec les conséquences douloureuses que cela emporte. En 2020, le Président de la République s'est engagé à mettre en place un plan de relance massif axé sur des secteurs d'avenir et sur les compétences, afin de bâtir notre souveraineté industrielle et écologique. Cette ambition s'est traduite par la présentation de la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné en France.

On peut citer l'étude Deplhy- déploiement de l'hydrogène en vallée de Seine -, qui cartographie l'ensemble des acteurs et des besoins actuels dans l'industrie et les mobilités lourdes

d'étendre notre souveraineté énergétique. Je souhaiterais donc savoir, madame la secrétaire d'État, ce que le Gouvernement entend faire pour accompagner les collectivités qui portent des projets de territoire au plus près des réalités locales. Comment comptez-vous favoriser ces prises d'initiative et inciter les élus locaux à s'emparer de ce sujet ?

qui a été lancé par l'Ademe le 14 octobre vise à soutenir dans les territoires le déploiement de projets importants d'infrastructures de production et de distribution d'hydrogène décarboné au regard des usages d'applications industrielles et de mobilité,

cette neutralité, l'hydrogène décarboné représente une véritable occasion d'accélérer la transition écologique tout en assurant l'indépendance énergétique de la France. Le 9 septembre dernier, le Gouvernement a présenté la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné. Un investissement de 7 milliards d'euros d'ici à 2030 est prévu, une enveloppe de 2 milliards d'euros étant déjà disponible dans le cadre du plan de relance. Nous ne pouvons que saluer ces financements indispensables pour accompagner les acteurs de l'hydrogène,

Des projets ambitieux voient le jour en France. En Vendée, l'entreprise Lhyfe, avec « hy » comme dans « hydrogène », a démarré un programme de construction de deux bâtiments dédiés à la production d'hydrogène vert par électrolyse et à la recherche-développement en matière de production d'hydrogène grâce à un parc éolien en mer

soutiendra et on accompagnera des investissements dans la production et la distribution d'hydrogène décarboné par des technologies ayant déjà fait l'objet de démonstrations et de premiers prédéploiements. Il s'agira prioritairement de projets orientés vers des usages industriels et la mobilité lourde, notamment dans le domaine des services publics et des transports lourds, collectifs ou de marchandises. Pour ce faire, des consortiums réunissant des autorités locales et des entreprises industrielles doivent travailler ensemble sur une même zone afin de créer ces écosystèmes à grande échelle, qui favorisent par ailleurs les économies d'échelle.

L'émergence de projets d'électrolyse raccordés directement à des installations d'énergie renouvelable est importante pour étudier les possibilités offertes par ce stockage de l'énergie.

l'hydrogène. Celui-ci est un vecteur de la transition énergétique ; il doit permettre de décarboner notre mix énergétique. Ce point ne semble pas contesté. Il ne fait aucun doute qu'il participera à l'indépendance énergétique de la France et à la stabilité de notre système électrique, grâce aux capacités de stockage À cela s'ajoutent les emplois directs et indirects qu'il créera, que l'on chiffre entre 50 000 et 100 000. Au-delà du cap économique, c'est le cap écologique qu'il nous faut plus que jamais tenir. Je pense aux objectifs fixés par l'accord de Paris, notamment à la réduction de 45 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et à la limitation à 1,5° de la hausse des températures d'ici à 2100 par rapport aux niveaux préindustriels. Cela suppose que 75 % du mix électrique soit produit à partir de sources faiblement émettrices à l'échelon mondial. À ce titre, l'essentiel se joue dans les dix années à venir : la décarbonation de l'ensemble des secteurs doit donc avancer à grands pas. À la question posée par notre débat, de savoir si la France peut devenir un champion de l'hydrogène, je répondrai : oui, mais il faut pour cela qu'elle s'associe à ses partenaires européens pour structurer et coordonner les investissements ; je pense en particulier aux réseaux La Commission européenne s'est également saisie du sujet en juillet dernier. Plusieurs États membres, tels que l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal, prennent les uns après les autres ce grand tournant avec des montants d'investissements proches des nôtres, voire plus ambitieux.

Si l'espoir existe, nous devons rester vigilants sur la bonne utilisation de la manne financière qui sera consacrée à l'hydrogène dans les prochaines années. Soutenir fortement un secteur pour constituer une filière est naturel et indispensable, mais un contrôle de l'efficacité des dépenses engagées est primordial.

en matière de recherche et développement, mais aussi de formation pour accompagner ces nouvelles compétences. La piste de l'hydrogène blanc, issu d'émanations d'hydrogène naturel depuis l'écorce terrestre, n'est pas évoquée dans la stratégie française, à l'inverse de celle qu'a adoptée l'Allemagne.